l’intention de faire disparaître les départements était bien réelle. Mais les gouvernements de gauche durent y renoncer devant l’évidence : les départements sont l’échelon adéquat pour concilier proximité et expertise dans l’exercice de leur cœur de compétences, à savoir les politiques sociales. ! Les Français, eux, l’avaient bien compris. Les mauvaises intentions durent céder devant la mobilisation… Devant ce premier échec, le mot d’ordre a été de « dévitaliser » les départements, employé par notre ancien collègue André Vallini, alors secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale. Un organe est dévitalisé quand on lui coupe son arrivée de sang artériel. Il en est de même pour une collectivité, quand on lui enlève ses ressources financières. Ce que n’a pas réussi à faire l’exécutif en 2016, Emmanuel Macron y est parvenu, par un effet différé de la suppression de la taxe d’habitation – elle même bombe à fragmentation démagogique qui, non contente de supprimer tout lien financier entre l’usager des services municipaux et la gouvernance municipale, alourdit chaque année de plus de 20 milliards d’euros la dette de l’État. Mais revenons aux départements : pour compenser la perte de taxe d’habitation des communes, il fut décidé d’attribuer à celles ci une part du foncier départemental, parachevant la dévitalisation annoncée. Cette décision fut prise à la suite de la publication d’un rapport cosigné par notre ex collègue Alain Richard, lequel regretta ensuite publiquement, me semble t il, que les départements se trouvent dépourvus de tout pouvoir de taux. Comprenne qui pourra ! Les départements n’ont plus de pouvoir de taux, donc plus de maîtrise de leurs recettes.

tout en imposant une baisse de 40 % de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements. Dévitalisation, vous disais je… La situation, nous la connaissons tous : les départements sont totalement dépendants du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), autrement dit de la situation du marché de l’occasion des logements. Et que l’on n’objecte pas que, sur cette recette, il y a un pouvoir de taux : la quasi totalité des départements applique le taux plafond, faute de pouvoir faire autrement. Alors que les départements ne peuvent désormais plus que constater leurs niveaux de recettes, ils voient les gouvernements successifs leur imposer leurs dépenses.

effondrement de la construction neuve et retrait du marché de la location des passoires thermiques, retrait non anticipé et mal accompagné. Dans cette crise du logement, à part la hausse des taux d’intérêt, le Gouvernement porte de lourdes responsabilités

En 2023 par rapport à 2022, l’épargne nette des départements aura baissé de 51,3 %, quand celle des communes aura progressé de 16,9 %, et la trésorerie brute des départements aura fléchi de 26,7 %, quand celle des communes n’aura diminué que de 2,7 %.

Pourtant, les départements se montrent solidaires entre eux, avec une péréquation forte et volontaire ; mais cela ne suffit plus. Devant le terrible effet de ciseaux que je viens de décrire, l’investissement et l’aide aux communes deviennent la variable d’ajustement. C’est consternant, parce que le département n’est pas que la collectivité du social : il joue un rôle de péréquation, de soutien aux communes, et d’équilibre entre le rural et l’urbain, dans des domaines tels que les routes, la fibre optique, les collèges, dont nous avons plus que jamais besoin.

quelle hypothèse de recettes de DMTO retenez vous pour 2024 ? Ensuite, quelle hypothèse d’évolution des trois allocations individuelles de solidarité et de l’aide sociale à l’enfance retenez vous pour cette même année, en sachant que les dépenses sociales représentent plus de 60 % – jusqu’à 68 % parfois – des dépenses de fonctionnement des départements ?

Mais peut être cela n’est il pas totalement étranger au fait que les électeurs départementaux ont le mauvais goût de confier leur destin très majoritairement à des gouvernances de droite et du centre… Monsieur le ministre, je conçois que cela puisse être agaçant ; faut il pour autant avancer dans la voie de la démolition de notre pays ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner l’opportunité de m’exprimer sur le sujet des finances des départements, dans un contexte, vous le savez, particulier pour nos finances publiques et pour nos départements. Dans la période que nous connaissons, les départements font en effet face, vous l’avez dit, monsieur le sénateur, à une inflexion certaine de leur situation financière, ce qui les place d’ailleurs dans une situation singulière par rapport aux autres niveaux de collectivité. D’un côté, les dépenses sont dynamiques, notamment les dépenses de fonctionnement, plus particulièrement celles de personnel, qui augmentent de 7,2 % ; il est vrai que les départements, comme l’État et les autres collectivités, sont concernés non seulement par la revalorisation du point d’indice, des salaires du personnel médico social, mais aussi

Au total, les recettes réelles de fonctionnement sont en baisse : c’est une spécificité propre à l’échelon départemental. Bien que ces chiffres ne soient pas définitifs et que la situation soit bien sûr hétérogène entre départements, l’État est particulièrement attentif à une telle inflexion. Dans ce cadre, je prends un premier engagement : celui de poursuivre un dialogue constant avec Départements de France et son président, François Sauvadet. Plusieurs rendez vous ont déjà été fixés : dès ce mois ci, puis en mai, lors de la publication définitive des comptes de nos départements, et de nouveau à l’automne, au mois de septembre ou d’octobre. En parallèle, quinze départements appellent une attention particulière, car ils sont susceptibles d’être les plus affectés. Soyez certains que nous sommes et resterons vigilants. Je me tiens d’ailleurs à la disposition des présidents de département qui souhaiteraient me rencontrer ; certains d’entre eux m’ont déjà sollicité.

Si les recettes de DMTO sont mises en avant, elles restent une part minoritaire de l’ensemble des recettes et se maintiennent à un niveau supérieur à celui de 2019, qui fut une très bonne année en la matière. Pour autant, il faut pouvoir soutenir les départements confrontés à des difficultés conjoncturelles en matière de perception de ces prélèvements. Grâce au mécanisme de péréquation, l’écart de recettes par habitant entre le département le mieux loti et celui qui l’est le moins bien diminue de 40 %. S’ajoute une mise en réserve des sommes non distribuées au titre de la péréquation, pour un montant de près de 250 millions d’euros à la fin de l’année 2023. En plus de cette péréquation, nous avons mis en place un fonds de sauvegarde des départements. Ce fonds de sauvegarde bénéficie d’abord aux collectivités confrontées à une baisse importante du produit des DMTO et touchées par une hausse significative des dépenses liées au revenu de solidarité active,

pour le fixer à 106 millions d’euros, grâce à un abondement de l’État, qui y contribue ainsi à parité avec les départements. Cet effort supplémentaire bénéficiera à quatorze départements dès cette année. dès cette année. Par exemple, la Gironde bénéficiera de 9 millions d’euros, le Val de Marne, de 7 millions d’euros ; ce sont des montants non négligeables. Toujours en matière de DMTO, il existe depuis 2022 un mécanisme d’assurance individuelle, qui autorise les départements à mettre en réserve une fraction de leur produit de DMTO après délibération. Au 31 janvier 2024, 35 départements avaient mis en réserve un total de 1 milliard d’euros. Je tiens ici à saluer ces 35 départements, qui ont pris leurs responsabilités face au caractère cyclique cyclique des recettes départementales assises sur l’évolution des prix de l’immobilier. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, dans une conjoncture difficile liée à des facteurs exogènes, comme le ralentissement du marché immobilier, les mécanismes protecteurs existent et l’État est au rendez vous.

de mieux couvrir les dépenses d’aide à l’autonomie des départements. Face à l’enjeu que représente la prise en charge des mineurs non accompagnés, là aussi l’État accompagne les départements, en augmentant de moitié son soutien budgétaire à ce titre, pour lui faire atteindre près de 100 millions d’euros en 2024. Dans cette période d’inflexion pour les finances des départements, la question des recettes est, je le sais, particulièrement sensible. J’ai évoqué la situation des DMTO et les mécanismes à l’œuvre pour amortir les effets de leur contraction.

de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) qui leur est affecté a crû de près de 7 % en 2023. C’est aussi ce qui permet d’amortir le recul des DMTO. Surtout, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2020 a introduit un mécanisme de versement d’une fraction de TVA supplémentaire, d’un montant de 250 millions d’euros, à destination des départements exposés à un reste à charge au titre des allocations de solidarité. Il s’agit là d’un levier supplémentaire pour soutenir les départements en difficulté. Enfin, je veux dire un mot plus général du contexte dans lequel s’inscrit la situation des départements.

Le premier allié de nos finances publiques est la croissance et, avec elle, l’activité et l’emploi. Or le contexte international et européen est incertain et peu favorable, marqué par la poursuite des chocs géopolitiques au Moyen Orient et en mer Rouge, de la guerre en Ukraine et par le ralentissement de l’activité chez nos partenaires européens. Nous avons dû, comme d’autres pays partenaires, vous le savez, revoir nos prévisions de croissance pour 2024. Nous faisons face à des prévisions de recettes en baisse, ce qui nous a conduits à prendre la décision d’annuler 10 milliards d’euros dans le budget de l’État. Ces annulations nécessitent un effort de tous les ministères sur l’ensemble de leurs dépenses de fonctionnement, sur la maîtrise de la masse salariale, sur le décalage d’un certain nombre de projets. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, l’État prend sa part dans les efforts consentis pour le redressement de nos finances publiques. les sénateurs, et je terminerai ainsi mon propos, j’en appelle à une responsabilité partagée : tout doit être mis en œuvre pour assurer le respect de notre trajectoire de finances publiques, notamment sur les dépenses de fonctionnement. Il serait temps ! Je sais que les élus locaux, dans leur immense majorité, partagent cet esprit de responsabilité. Nous avons tous les finances publiques

équivalente. Il aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.

100 millions d’euros ou 30 %, c’est ce que représente pour le département dont je suis élue, l’Essonne, la diminution du montant des droits de mutation à titre onéreux en 2023. À l’échelle nationale, les départements auront perdu 3,9 milliards d’euros entre 2022 et 2023. relatives aux allocations individuelles de solidarité – APA, PCH et RSA – pèsent pour plus de 18 milliards d’euros, avec un reste à charge de 50 % pour nos collectivités. Songez également que les dépenses au titre de l’aide sociale à l’enfance représentent, à elles seules, près de 10 milliards d’euros. Les départements doivent en outre assumer les conséquences d’une politique migratoire hors de contrôle, avec notamment l’arrivée de mineurs non accompagnés. La prise en charge de ces derniers leur coûte plus de 2 milliards d’euros, avec une compensation de 6 % seulement. Leur situation financière est devenue d’autant plus critique que les dépenses supplémentaires imposées par l’État, soit 2,5 milliards d’euros de plus en deux ans, n’ont, une fois encore, pas été compensées. Jusqu’à présent, vous aviez beau jeu de dire que, pour faire face à ces dépenses nouvelles, les départements pouvaient s’appuyer sur leurs recettes de DMTO supplémentaires, devenues stratégiques. Mais, aujourd’hui, ces dernières ont disparu et les recettes sont revenues à leur niveau d’avant covid, alors que les dépenses, elles, subsistent. la crise des finances départementales n’est pas une vue de l’esprit. Depuis la réforme de la taxe d’habitation, les départements ne disposent plus de levier en matière de fiscalité. L’investissement et l’aide aux communes ne doivent pas devenir la variable d’ajustement de leurs budgets. mènent en effet des politiques volontaristes de péréquation et d’équilibre entre le monde rural et les territoires urbains. Nous ne voulons pas renoncer à ces politiques vertueuses par nécessité budgétaire. Oui, nos départements revendiquent une autonomie fiscale pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le législateur. Monsieur le ministre, ma question est la suivante : quand le Gouvernement va t il enfin prendre la mesure de la gravité de la situation et déterminer un panier de ressources permettant aux départements de faire face à leurs charges, comme le demande depuis longtemps le Sénat ? La parole est à M. le ministre délégué. Madame la sénatrice,

conséquence de l’inflation soutenue, de la revalorisation du point d’indice, de la chute des recettes de DMTO, de l’insuffisance de la compensation des allocations individuelles de solidarité, des dépenses imprévues, comme celles qui sont liées à l’accueil des MNA, et ce en l’absence, contrairement à ce que je viens d’entendre, de toute autonomie fiscale et même financière financière des départements. Je souhaite vous interroger tout particulièrement sur les dépenses de personnel. Chacun le sait, l’augmentation du point d’indice ne dépend en aucun cas de la volonté des collectivités locales ; c’est l’État qui la fixe. Les revalorisations sectorielles définies dans le cadre du Ségur de la santé, même si elles ne sont pas contestables, altèrent fortement le niveau des dépenses de personnel. L’ajustement des régimes indemnitaires et des avantages sociaux, mis en œuvre pour conserver l’attractivité des employeurs publics, dans un contexte de crise sur le marché de l’emploi, mine également les collectivités locales que sont les départements. départements. Monsieur le ministre, comment le Gouvernement compte t il accompagner les départements, notamment lorsque c’est l’État qui décide de rehausser fortement le point d’indice sans concertation avec les collectivités locales ? J’évoquerai un second point, le financement de la protection civile, qui devient évidemment essentiel dans un contexte où les départements et les territoires, notamment de montagne, sont exposés aux aléas climatiques. Des négociations sont actuellement menées à l’échelon européen à propos du statut des sapeurs pompiers volontaires, qui pourraient être assimilés à des salariés de droit commun.

sur le point d’indice et le financement de la protection civile. Sur le point d’indice, il n’aurait pas été, à mon sens, responsable de ne pas proposer aux agents publics de mesures face au choc inflationniste que nous avons rencontré.

milliard d’euros en 2023, contre 900 millions d’euros initialement. En dix ans, cette fraction a augmenté de plus de 36 %. Le département des Hautes Alpes a ainsi perçu plus de 3 millions d’euros, contre 2 millions d’euros dix ans plus tôt. À l’occasion du débat sur le projet de loi de finances,

est à M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, regarder la situation des départements, ce n’est pas uniquement s’intéresser à l’effet de ciseaux financier actuel ou à la fiscalité, c’est aussi, comme l’évoquait mon collègue précédemment, considérer la pente des dépenses. De ce point de vue, je veux, pour illustrer mon propos, m’arrêter sur la protection de l’enfance. Le nombre des mesures engagées au titre des enfants placés à l’échelle nationale a quasi doublé en vingt ans, avec une accélération brutale depuis 2019.

chaque année de la branche famille de la CAF, notamment en matière de prévention sur le terrain

mais l’article 72 2 de la Constitution est balayé par cette affectation d’une fraction de la TVA ; c’est la fin de l’autonomie ! La démocratie locale s’en trouve altérée et menacée. Les services publics départementaux constituent encore le premier levier de la redistribution, le plus fidèle soutien des communes et le meilleur outil de cohésion territoriale.

Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, c’est un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, ce n’est pas une proposition du Gouvernement ! Oh, pardon… Je vous l’affirme, il n’y a pas de projet de suppression des droits de mutation à titre onéreux : j’espère que cela vous

Qu’est ce qui garantit la libre administration des collectivités territoriales ? C’est l’autonomie financière, c’est à dire par la capacité d’avoir des ressources et de les employer librement. Pas toujours ! L’autonomie fiscale, c’est la capacité de moduler le taux d’un impôt. Mais au service de quel projet ?

L’effet de ciseaux tant décrié par les départements est devenu une constante budgétaire et chaque nouvelle annonce alourdit un peu plus cet effet « de sécateur

Sans autonomie fiscale, l’impossibilité de prévoir ces coûts pour les collectivités se traduira par un recul de l’investissement public, pourtant au cœur des missions des départements en faveur de la solidarité territoriale. Monsieur le ministre, vous connaissez le rôle de pilier que jouent les départements dans notre équilibre institutionnel. Le moment n’est il pas venu, alors qu’une mission sur la décentralisation est en cours, d’instaurer

Par ailleurs, le montant global des dépenses en matière d’action sociale varie également selon les collectivités. Ces deux facteurs expliquent pourquoi certains départements se portent financièrement moins bien

en 2022 des résultats globalement favorables. Les évolutions positives des recettes de fonctionnement et l’augmentation du point d’indice ont permis à l’épargne brute des départements de croître de 5,3

cousue main. J’ai toujours défendu cette idée : n’ayons pas une vision homogène des collectivités territoriales, car nos territoires sont tous différents, vous êtes bien placés pour le savoir,

de la baisse des DMTO, de l’augmentation des charges de personnels et des dépenses sociales, cette décision met en péril l’équilibre budgétaire déjà fragile de nos départements. Le basculement des 320 000 bénéficiaires de l’ASS vers le RSA coûterait plus de 2 milliards d’euros

Comptez sur notre détermination à travailler avec les départements pour mieux accompagner les bénéficiaires du RSA et limiter les dépenses des départements au titre de cette politique. La parole est à Mme Briquet, pour la réplique. Monsieur le ministre, je crains de ne pas partager votre optimisme. Je ne crois pas à l’emploi magique. Au delà du problème financier, votre réforme provoquera une réduction des droits sociaux et la paupérisation de citoyens déjà fragiles.

Cette suppression revient à accroître la précarité pour bon nombre de nos concitoyens et pour nos départements. Mme Valérie Boyer. Monsieur le ministre, le nombre de MNA intégrant les dispositifs de protection de l’enfance a été pratiquement multiplié par quatre entre 2014 et 2023, passant de 5 000 à 19 370

en réalité aux collectivités départementales de gérer un problème qui relève du domaine régalien. L’association Départements de France tire donc la sonnette d’alarme, car la situation devient critique, pour ne pas dire dramatique. Les dispositifs de l’ASE, l’ASE, longs à se mettre en place, sont aujourd’hui menacés par cet afflux trop important et non maîtrisé. Est ce faire preuve d’humanité que d’enrichir toujours plus les filières mafieuses ou criminelles avec de tels trafics d’êtres humains ? Il est en effet clair que les MNA n’entrent jamais seuls,

Comment comptez vous aider les départements à mobiliser les 5,5 milliards d’euros nécessaires à ce transfert ?

le président de ce département, Stéphane Troussel. Nos départements sont confrontés à une hausse sans précédent de la demande sociale de la part de nos concitoyens. Pourtant, les réformes successives n’ont fait que réduire leurs marges de manœuvre financières et accroître la dépendance de leurs ressources à la conjoncture économique : gel des dotations de fonctionnement, transfert de la taxe foncière aux communes, suppression de la CVAE. Cette dépendance financière fragilise leur rôle d’amortisseur de crises, lequel devrait plutôt conduire l’État à les doter d’une structure financière stable et solide. 2023 illustre la fragilité des budgets départementaux, en raison de la chute généralisée et sans précédent des droits de mutation, pour près d’un quart entre 2022 et 2023. Les situations sont beaucoup plus dégradées

Dans ce contexte, plusieurs départements ont dû fortement réduire leurs investissements pour 2024 et les années suivantes. Pourtant, les collectivités territoriales jouent un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Elles devront investir au moins 12 milliards d’euros par an à l’horizon de 2030, soit le double de ce qu’elles dépensent actuellement. Pour la seule rénovation thermique de leurs bâtiments, les besoins sont colossaux, de l’ordre de 3 milliards d’euros par an. Afin de faire face à ce mur d’investissement, l’État a certes mis en place le fonds vert, qui permet d’apporter un financement complémentaire à certains projets, mais les élus départementaux ne peuvent que constater

insoluble. Alors qu’en raison de leurs compétences les départements sont en première ligne pour affronter les grands défis sociaux de notre époque, ils doivent aussi être en mesure d’accélérer drastiquement leurs investissements en matière de transition écologique. Comment comptez vous les aider structurellement à répondre à ces impératifs de société ?

d’un consensus plein et entier dans cet hémicycle –, l’autonomie financière des collectivités territoriales, et singulièrement des départements, a progressé.

soit il est temps d’avouer qu’il s’agit d’une stratégie visant à faire des départements de simples opérateurs de l’État, en faisant fi du principe de libre administration des collectivités ; soit il faut urgemment redonner des marges de manœuvre et une salutaire capacité d’agir à cet échelon départemental, au profit des solidarités humaines et de l’équilibre des territoires.

Puisque vous aimez cette expression, monsieur le ministre, permettez moi, avec Mme Espagnac, sénatrice des Pyrénées Atlantiques, de vous inviter à un voyage, à un voyage d’Évry à Biarritz, un voyage non pas pour découvrir les charmes et les richesses du patrimoine de nos deux départements, mais un voyage pour vous montrer à quel point les problématiques de terrain sont identiques et prégnantes dans des territoires pourtant différents. Ainsi, les ex bénéficiaires de l’ASS vont, dès 2025, se retrouver dans une situation de précarité intenable. Ils devront alors se tourner légitimement vers les aides potentielles des départements.

Monsieur le ministre, le Gouvernement va t il participer et compenser tout ou partie des pertes de ressources des départements et participer à l’effort de solidarité ? Sinon, comment envisager que les départements puissent investir dans la transition écologique, sur le réseau routier ou dans les équipements destinés aux pompiers ?

puisque vous nous donnez l’impression, chaque fois, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ce qui laisse dubitatifs un certain nombre d’élus départementaux. En effet, la réalité est bien différente. Beaucoup de mes collègues l’ont déjà décrite. Votre « cousu main », monsieur le ministre, a un petit arrière goût de tutelle de l’État sur les collectivités locales. En cette période de, permettez moi d’observer que le corset imposé aux départements est bien trop serré et qu’il étouffe le budget de nos collectivités. Laissez les donc respirer

la suppression de tout lien fiscal avec nos administrés, à la suite de la perte du foncier bâti, remplacé par une dépendance à des dotations d’État plafonnées, non indexées sur l’inflation. Nous n’avons plus aucune marge de manœuvre et nous prenons de plein fouet l’effondrement du marché de l’immobilier. Vous ne pourrez plus, monsieur le ministre, parler d’autonomie financière ; j’ose du l’augmentation de la rémunération du personnel – sans concertation préalable –, la hausse du RSA et les revalorisations dans le médico social – sans vision de long terme – détruisent nos capacités financières. Bientôt, la solidarité à la source et la fin de l’allocation de solidarité spécifique nous achèveront. Dans le même temps, nous subissons l’explosion de nos dépenses sociales liées à la montée des précarités. Les Ehpad sont en difficulté, la protection de l’enfance sature et nous devons faire face à la hausse des flux migratoires, avec l’accueil des mineurs non accompagnés. Ici même, devant la délégation aux collectivités le président de l’Assemblée des départements de France, M. François Sauvadet, a parlé d’une véritable asphyxie, avec des conséquences désastreuses sur l’aide au monde rural et sur les communes. Ce constat, que vous connaissez et que donc vous assumez, est analysé par beaucoup comme une condamnation à mort des départements. Ma question, monsieur le ministre, est donc simple : souhaitez vous contredire ces affirmations ?

créant ainsi une disparité dans la gestion de cette ressource vitale. Cette technicité et la perte de compétences engendrent un écart entre les ambitions d’une gestion démocratique de l’eau et la réalité.

quelles aides financières précises le Gouvernement envisage t il de proposer pour soutenir les départements dans leurs projets de politique de l’eau, afin qu’ils assurent une gestion durable et équilibrée de cette ressource essentielle, tout en surmontant les obstacles juridiques actuels ?

que les départements recherchent un certain nombre de produits fiscaux. Dans la Loire, département dont je suis élu, lors d’une enquête menée auprès des communes, 84 % des maires ont répondu que leurs projets d’aménagement ou de développement de services

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite de la tenue de ce débat qui, j’espère, permettra des avancées concrètes. S’il y a un enseignement qui se dégage de débat, et qui sans doute était déjà établi, c’est bien celui d’un consensus quant à la situation financière des départements. Ils sont le niveau de collectivité dont la situation est la plus dégradée, car le plus exposé à la conjoncture, mais pas seulement, comme nous allons le voir. Lors de l’examen du budget de 2024, vous aviez d’ailleurs admis cette situation et vous vous étiez engagé à traiter cette question sans délai. Nous y voilà donc. En effet, les réponses apportées lors de l’examen du budget étaient très largement insuffisantes, pour ne pas dire indigentes. Elles consistaient pour l’essentiel à maintenir à flot ceux qui risquaient de se noyer, et encore… Rappelons tout d’abord que les départements ont été vertueux et solidaires. C’est le seul niveau de collectivité qui a organisé une péréquation horizontale, dont vous avez d’ailleurs permis l’amplification, qui a eu une approche collective et qui a instauré des mises en réserve.

sur les deux dernières années, l’augmentation des dépenses des départements non compensée par l’État s’élève à 2,5 milliards d’euros, en raison notamment de décisions du Gouvernement qui se sont imposées aux départements, telles que la revalorisation du point d’indice ou de certaines prestations sociales. Plus spécifiquement, sur les dépenses sociales, les départements subiront une nouvelle hausse du RSA, qui représentera 460 millions d’euros en 2024 – au passage, je conteste le chiffre de 97,5 % de couverture que vous avez avancé précédemment, monsieur le ministre –, un reste un reste à charge des AIS qui s’élève à plus de 9 milliards d’euros et représente désormais plus de 50 % de la dépense, une explosion des dépenses de l’aide sociale à l’enfance, qui atteindront 10 milliards d’euros soit une hausse de près d’un tiers en dix ans,

Comme toutes les collectivités, les départements ont également été – et le sont encore, bien sûr – confrontés à l’inflation. Ils ne sont pas que les collectivités du social, même si ce secteur représente, avec le médico social, 68 % de leurs dépenses de fonctionnement

Cet effet de ciseaux n’est plus soutenable et met en cause les missions essentielles de cette collectivité de proximité et de bonne dimension. C’est un amortisseur social, mais aussi territorial, même si cet aspect a été amoindri par la loi NOTRe, qui devra en outre faire face à un choc démographique que nous savons inéluctable et qui engendrera une hausse des dépenses liées à la prise en charge des personnes âgées, comme on le voit déjà dans les Ehpad. Plus encore, l’asphyxie des départements fait courir un véritable risque à notre modèle de décentralisation, auquel je suis, comme vous tous, très attaché et que je voudrais voir amplifié plutôt que rogné sans cesse. Le Sénat a fait des propositions en ce sens, sans attendre la mission Woerth, à laquelle il contribue également. À cet égard, la recentralisation pérenne du RSA dans trois départements ou à titre d’expérimentation – en Seine Saint Denis, dans les Pyrénées Orientales et dans l’Ariège – ne me paraît pas de

nos concitoyens. Je veux insister sur la nécessité de revoir en profondeur le système de financement des départements, dont les ressources principales, les DMTO, évoluent de manière contradictoire avec leurs dépenses. En effet, les départements sont essentiellement financés par les DMTO dépendant largement de

sur les finances des départements. Mes chers collègues, en raison du nombre d’amendements déposés sur la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, nous pourrions siéger jeudi 7 mars après midi et, éventuellement, le soir. Y a t il des observations ?…

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre débat porte sur le sujet suivant : la France est elle prête pour accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques, les JOP, événement populaire qui sera la plus grande fête du sport jamais organisée en France une occasion unique de mettre en avant notre pays, qui sera sous le feu des projecteurs mondiaux. On estime à 4 milliards le nombre de téléspectateurs qui visionneront les JOP, soit la moitié de l’humanité Si ces chiffres sont certes enthousiasmants, ils nous obligent à veiller à ce que cette grande fête du sport se réalise dans les meilleures conditions possible. La France a une longue histoire d’accueil des plus grands événements sportifs internationaux. L’organisation des JOP de Paris 2024 marquera le point d’orgue de ce savoir faire français, qui rayonnera à l’étranger et sera utile dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, qui se dérouleront en Auvergne Rhône Alpes et en région Sud.

Il faut saluer également le travail des différents ministères, des services de l’État et des collectivités territoriales, qui remplissent des missions primordiales comme la sécurité ou encore l’organisation des transports et les multiples missions de logistique. Malgré tout cela, certaines interrogations subsistent ou prennent forme à la veille de cet événement mondial. Revenons dans un premier temps sur le travail de la Solideo, qui, depuis l’annonce de ses ambitions en 2018, réussira à livrer dans les temps les ouvrages nécessaires aux JOP.

Pour les ouvrages prévus pour la phase « héritage », au moins quatre des huit piscines neuves ou rénovées ont été livrées ou sont en passe de l’être. Le coût total des ouvrages nécessaires aux jeux avait été évalué à 3,8 milliards d’euros. Le budget, il faut le souligner, devrait être maîtrisé. Nous pouvons saluer le travail de la Solideo, qui devrait réussir à répondre fidèlement à un cahier des charges ambitieux sur les plans environnemental et urbanistique. Je note cependant deux points de vigilance, à savoir les chantiers du Grand Palais éphémère pour les épreuves de judo et de lutte, dont le calendrier est extrêmement serré, ainsi que la piscine de Colombes, qui accueillera les entraînements pour la natation synchronisée et devrait être livrée au début du mois de juin. Le directeur général de la Solideo nous a assurés, lors de son audition en janvier dernier, que ces chantiers devraient être livrés à temps. concerne les transports, plusieurs facteurs risquent de perturber le bon déroulement des Jeux. Tout d’abord, nous constatons dès à présent que la situation dégradée du trafic dans les transports en commun reste problématique. Nous n’avons pas encore retrouvé le niveau de service d’avant covid. Au mois d’août prochain, avec les Jeux, le trafic sera classique, avec 15 % d’activité en plus, alors que, normalement, à cette période, le trafic baisse de 30 % à 40 %. Cette hausse d’activité suscite de vraies inquiétudes, tout comme le recrutement des agents, qui n’est pas encore, à l’heure actuelle,

dans la réalité, un syndicat a déposé voilà un mois un préavis de grève englobant l’ensemble de la période des Jeux. Nous l’avons bien compris, le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, de réformer le droit de grève. Pourtant, l’image de notre pays serait largement écornée, voire ridiculisée, si nous devions voir nos services de transports publics ou de ramassage d’ordures gelés en plein Avec un délai de prévenance inexistant, la possibilité de préavis de grève à durée illimitée est réelle. Qu’avez vous prévu, madame la ministre, pour garantir le bon fonctionnement des services publics et préserver l’image de la France ? l’offre de transport, hormis la mise en service du prolongement de la ligne 14 à Paris, il faudra faire en Île de France avec les infrastructures et le matériel vieillissant existants. Le Cojop prévoit des navettes, notamment pour le transport des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, ces services seront temporaires et sont prévus pour la durée des Jeux, sans héritage pour la population francilienne ; c’est une occasion manquée. Si nous comprenons la difficulté de rendre accessible l’ensemble du réseau, il serait intéressant de disposer d’un engagement sur la rénovation de chaque station de métro, afin que l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite soit systématiquement prise en compte. Cela contribuerait à l’héritage des Jeux et enclencherait une stratégie d’amélioration continue. nous saluons les efforts consentis, notamment par la région Île de France, dont l’objectif est de former 15 000 personnes aux métiers de l’accueil et de la sécurité, pour garantir la bonne tenue des jeux Olympiques. Mais les efforts de la région doivent être accompagnés pour être suffisants, pour assurer une meilleure sécurité. Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques nous a confirmé le défi de mobilisation que représente le recrutement des agents de sécurité privée qui compléteront les effectifs de police et gendarmerie.

Le soutien à nos athlètes ne doit pas s’arrêter à la clôture des Jeux. La récente annonce de l’annulation de 50,5 millions d’euros de crédits destinés au ministère des sports a de quoi nous inquiéter. Pourtant, madame la ministre, vous aviez beaucoup communiqué, à l’automne dernier, sur l’augmentation de ses crédits. Or la réduction annoncée annule tout simplement la hausse

Ces baisses s’inscrivent dans une tendance plus large de diminution des crédits pour le sport, qui pourrait représenter 130 millions d’euros sur 2025 et 2026. Permettez moi de m’inquiéter de la stabilité à long terme des financements pour le sport. Pour conclure, je souhaite féliciter une nouvelle fois l’ensemble des acteurs impliqués dans la réussite de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il nous reste 143 jours pour accompagner l’ensemble des acteurs et pour livrer des JOP historiques pour notre pays. Soyons tous à la hauteur de cet enjeu, qui ne doit pas s’arrêter le jour de la clôture des Jeux, mais perdurer, afin que notre pays bénéficie des retombées sociales et économiques de cet événement, dans lequel nous avons beaucoup investi. Nous attendons tous un succès de l’organisation des Jeux et de nombreuses médailles, mais le plus grand succès sera avant tout celui de l’augmentation de la pratique sportive par nos compatriotes, afin que notre pays soit enfin une nation sportive.

et les plus responsables de l’histoire. Comme j’ai coutume de dire, il y a quatre dimensions dans la réussite des jeux : l’organisation, la performance des athlètes, l’engagement et l’héritage. En ce qui concerne l’organisation, nous sommes dans nos « temps de passage » pour la livraison de Jeux exemplaires. Vous l’avez dit, la Solideo est en train de réussir l’exploit de bâtir l’ensemble des infrastructures dans le respect des meilleures exigences sociales et environnementales, tout en respectant le calendrier et et le budget : c’est une première dans l’histoire des Jeux et une immense réussite pour notre pays, nation de bâtisseurs. Nous pouvons en être fiers Après la livraison de l’Arena Porte de la Chapelle et du village des athlètes la semaine dernière, le village des médias et le centre aquatique olympique seront à leur tour inaugurés, respectivement le 25 mars et le 4 avril

porte ses fruits, avec 16 700 entrées en formation et plus de 10 000 recrutements sécurisés ; les plans de mobilisation de nos forces de l’ordre sont calés ; et la préparation de la cérémonie d’ouverture fait l’objet d’un suivi particulier. restriction de circulation définitifs ont été présentés par le préfet de police le 1 mars dernier, pour l’Île de France, permettant aux riverains et aux acteurs économiques d’anticiper les impacts.

en moyenne, de 15 % et, si nécessaire, jusqu’à 60 %. Nos grands chantiers d’infrastructures sont également parfaitement dans les temps, comme en atteste le lancement réussi du nouveau système de pilotage automatisé de la ligne 14, qui sera la colonne vertébrale de la desserte des jeux. Le dialogue social se poursuit dans le cadre des plans de maintien d’activité des administrations publiques, tout comme celui qui est mené en autonomie par les opérateurs de transports Nous faisons en sorte que les sujétions spécifiques auxquelles les équipes seront exposées à l’été 2024 soient dûment prises en compte. J’ai pleinement confiance dans l’esprit de responsabilité de chacun, pour valoriser la mobilisation exceptionnelle

et des opérateurs de transport, l’État prend toute sa part, le cofinancement de la mise en accessibilité des cheminements entre les gares et les sites et la mise en place d’un fonds de 300 millions d’euros, dont 100 millions d’euros seront fléchés prioritairement vers les hôtels, restaurants et petits commerces des villes accueillant les Jeux, dès l’exercice 2024. Sur les enjeux sanitaires, nous sommes au travail avec les ministres compétents pour que notre système de santé réponde pleinement

Les Jeux sont aussi une occasion unique de renforcer la qualité de l’accueil touristique sur notre territoire et de promouvoir auprès des touristes du monde entier nos savoir faire faire : dès le relais de la flamme olympique seront organisés des programmes de tourisme industriel et des marchés de producteurs locaux, en même temps que nous mettrons en valeur de notre patrimoine au travers de plus de 400 villes françaises, y compris en outre mer. prêts, sur le plan diplomatique, à délivrer les 70 000 visas nécessaires à la famille olympique et à veiller au respect de la stricte neutralité des athlètes russes et biélorusses qui concourront,

les fédérations olympiques et paralympiques pour continuer à porter avec elle la bonne avancée opérationnelle de notre préparation dans l’ensemble des domaines, de l’antidopage à la gestion logistique de nos délégations. Sur le sujet de l’engagement, nous sommes prêts à déployer l’ensemble de nos dispositifs pour faire vivre à tous nos concitoyens une grande fête populaire. Je veux le rappeler, nos Jeux seront les plus décentralisés de l’histoire, avec 73 collectivités hôtes. Dans deux mois, le relais de la flamme marquera le coup d’envoi de l’aventure olympique et traversera près de 70 départements de notre pays. Sur le terrain, j’ai pu encore le mesurer ce matin dans l’Yonne, les acteurs et les élus locaux programment l’ensemble de leurs festivités autour du relais, en complémentarité avec l’Olympiade culturelle culturelle et la programmation sportive de la grande cause nationale, qui fait l’objet de plans d’action territoriaux soutenus à hauteur de 4 millions d’euros par mon ministère. concerne les zones de célébration pendant les Jeux, les clubs 2024, plus de 250 projets ont été déposés par les collectivités et doivent maintenant être validés par les préfets, avec pour objectif la meilleure couverture possible de nos territoires et un principe de sécurisation par des moyens exclusivement locaux. Dans le même objectif de mobilisation de tous les Français, les prochaines semaines : la Semaine olympique et paralympique, la SOP, ainsi que le plan Été olympique et paralympique, pour faire vivre un été exceptionnel de sport à notre jeunesse, avec des séjours, des découvertes et des animations sportives

offre 400 000 places, dont 200 000 pour le public scolaire en provenance de toutes les académies de notre pays. Enfin, pour ce qui a trait à l’héritage, nous sommes prêts à léguer à notre pays

des athlètes au franchissement urbain Pleyel, le FUP, les différentes opérations d’aménagement nous permettent de « recoudre » le territoire de la Seine Saint Denis. Le FUP sera inauguré dans les toutes prochaines semaines, et nous léguerons 19 bassins

et au développement du sport santé dans l’ensemble de nos territoires, au diapason de notre grande cause nationale ! Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avançons vite et bien. Je compte sur vous pour être, avec nous, les ambassadeurs de cette mobilisation collective au service de la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons

ont vocation à servir cette ambition, l’atteinte d’un tel objectif suppose la mise en œuvre d’un cadre logistique d’accueil éprouvé, afin d’assurer, entre autres, la sécurité et le transport des 15 millions de visiteurs qui s’apprêtent à converger vers le territoire francilien et les différentes villes hôtes. La construction de ce cadre est aujourd’hui en partie assurée par les acteurs de l’industrie des événements professionnels, qui mettent au profit des jeux toute l’expertise et le savoir faire que l’organisation répétée d’événements d’envergure internationale leur confère. Un héritage durable est devenu la condition essentielle de l’acceptabilité des JOP par l’ensemble des professionnels mobilisés sur cet événement, mais aussi par l’ensemble des Français concernés. Or une part essentielle de cet héritage est pourtant négligée. Il s’agit de son volet socioéconomique, qui s’appuie notamment sur les dispositifs de soutien mis en œuvre par le Gouvernement pour accompagner les pratiques des professionnels concernés ayant vocation à rendre l’expérience des touristes sportifs inoubliable. Cette expérience client passe, entre autres, par un accueil amélioré aux frontières et par un parcours sécurisé des visiteurs après leur arrivée à destination. C’est cet héritage qui permettra à la France de rattraper le retard qu’elle accuse depuis plusieurs années dans l’accueil d’événements internationaux à d’autres destinations concurrentes. Nos voisins européens l’ont bien compris : dans ces pays, les acteurs publics et privés des secteurs concernés travaillent main dans la main pour assurer une haute qualité d’accueil et de séjour à leurs visiteurs, touristes et voyageurs d’affaires.

Au regard de cet éclairage, et étant entendu que je n’ai aucun doute sur la réussite des Jeux, quels sont, madame la ministre, les moyens mis en œuvre par le Gouvernement afin que cet héritage socioéconomique coconstruit avec les professionnels soit pérennisé au delà ? La parole

celui des EDE, les, qui nous permet de nous appuyer sur de grands acteurs de l’événementiel pour organiser nos opérations dans les différents sites de compétition. En outre, je m’assure, dans le cadre de l’action diplomatique de mon ministère, que nous aidons nos entreprises à faire rayonner leur savoir faire

précaires et mal rémunérés, ainsi que par des horaires très contraints. Le rendez vous étant présenté comme « à risque », le dispositif doit reposer sur des personnes qualifiées et professionnelles. Où en êtes vous de votre politique de recrutement et de formation de ces agents ? Je souhaite conclure en revenant sur le sujet de la compétition de surf de Tahiti.

Cet engagement repose sur un schéma national des mobilités, qui nous permettra d’organiser tous ces flux de transport à l’échelle du pays ; il sera publié, en lien avec les préfets et les collectivités concernées,

des spectateurs et des accrédités, qui justifie la mise en place des plans de transport que vous évoquez ; ensuite, minimiser les impacts sur le quotidien des autres usagers.

à s’exprimer, portant notamment sur les infrastructures dédiées aux JO. Seront elles en mesure d’accueillir les millions de spectateurs attendus ? Par ailleurs, en Île de France, où les transports sont déjà saturés et où la sécurité est une préoccupation constante, sommes nous prêts à gérer l’afflux de visiteurs et d’athlètes qui vont déferler sur notre région à l’occasion des jeux Olympiques ? Les transports représentent un défi colossal et, là encore, les inquiétudes sont nombreuses. On s’interroge sur les moyens qui seront mis en œuvre pour garantir une mobilité fluide pendant ces JO. Malgré la création de voies olympiques dédiées, le risque d’embouteillages d’une ampleur inédite en Île de France plane sur les Jeux. Enfin, la question de la sécurité se pose de manière constante. Madame la ministre, à cinq mois de la cérémonie d’ouverture, bien trop d’incertitudes persistent : comment pouvez vous rassurer les Français quant au bon déroulement de ces Jeux ? La parole est

du village olympique procurera aux habitants 3 000 logements, dont 45 % de logements sociaux, des groupes scolaires, des résidences étudiantes, carrés de bureaux et des commerces, tout cela parfaitement inséré dans le tissu des trois villes concernées. Nous léguons aussi à la Seine

qui est des transports, je l’ai dit, nous sommes mus par une double volonté de programmation et d’anticipation. Nous avons développé des infrastructures, dont la ligne 14, qui sera l’axe central de la desserte des Jeux,

en matière d’infrastructures. Au delà du village olympique, inauguré la semaine dernière par le Président de la République, pouvez vous nous indiquer, madame la ministre, quelles sont les infrastructures qu’il reste à bâtir, afin d’accueillir dans des conditions optimales les 10 500 athlètes internationaux ? Mes chers collègues, se demander si la France est prête pour ces JO, c’est également s’interroger sur leur héritage en matière de réutilisation des infrastructures. Or l’histoire démontre, hélas ! que l’héritage des infrastructures pose parfois des difficultés. Je pense aux fameux « éléphants blancs », ces infrastructures à l’envergure prestigieuse qui, au lendemain des Jeux, se révèlent en définitive plus coûteuses que bénéfiques et dont l’exploitation ou l’entretien devient un fardeau financier. Il en est de

construits entre les éditions d’Athènes, en 1896, et de Pyeongchang, en 2018, sont aujourd’hui utilisés, 11 % de ces sites n’existent plus et 4 % d’entre eux sont fermés, inactifs ou abandonnés. Madame la ministre, puisque les Jeux de Paris se veulent exemplaires, pouvez vous nous assurer qu’aucun éléphant blanc ne verra le jour ? Enfin, ces Jeux sont également, et doivent être, ceux de tous les Français, car de nombreux territoires accueilleront des entraînements et des compétitions sportives. Madame la ministre, dans quelle mesure tous les territoires concernés pourront ils eux aussi bénéficier de l’héritage des Jeux ? La

Nous avons à cœur, dans l’ensemble des territoires, d’utiliser et de mettre en valeur nos capacités sportives. Je pense aux près de mille centres de préparation aux Jeux qui verront les athlètes du monde entier s’entraîner au contact des populations. J’étais récemment

monter en puissance dans leur préparation et incarner les Jeux. Nous avons aussi à cœur, avec le relais de la flamme, la billetterie populaire,

Tony Estanguet affirmait, le 31 décembre dernier : « On sera prêts pour les Jeux. » Émanant du président du Cojop, des propos contraires eussent été inquiétants. La France attend cet événement depuis un siècle ; le spectacle du 26 juillet prochain devra être le prélude de Jeux réussis, dont nos compatriotes seront fiers. en être les ingrédients ? Une sécurité à toute épreuve ; soixante médailles françaises ; une exemplarité environnementale ; des Jeux socialement irréprochables ; un budget maîtrisé et transparent ; des équipements fonctionnels ; mais aussi des Jeux vraiment populaires, pierre de touche du succès de la compétition. D’où ma question : les conditions sont elles remplies pour faire de ces Jeux un événement impliquant le maximum de nos concitoyens et de nos territoires ? Mon interrogation porte également sur le sens

Enfin, sommes nous capables de faire des Jeux le catalyseur d’un projet sportif global plus ambitieux à l’horizon d’une vingtaine d’années, en termes d’emploi, de bénévolat, de sport scolaire ou d’enjeux sociétaux liés au handicap et à la sédentarité, au renforcement de la citoyenneté et à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence ?

pour les collectivités concernées et pour les départements qui ont fait l’effort de s’embarquer dans ce relais. La billetterie populaire va nous permettre d’emmener aux Jeux 400 000 personnes,

Cependant, depuis quelques mois, le rêve ne cesse de se confronter à la réalité, c’est à dire aux nombreuses inquiétudes que l’organisation de cette cérémonie suscite chez les Parisiens.

ambition. Le Président de la République l’a dit : en cas d’accroissement très fort de la menace, qu’elle soit terroriste ou d’une autre nature, nous serions bien évidemment conduits à activer un plan B, que nous préparons dans les conditions de confidentialité requises. La parole

plus particulièrement pour les Parisiens, dont le quotidien sera plus que jamais rythmé et affecté par cet événement exceptionnel. Nous appelons le Gouvernement à la plus grande vigilance, car c’est l’image de la France qui est en jeu.

je souhaite vous parler de la sécurité civile, celle qui consistera à lutter contre les incendies ou à gérer les accidents et qui sera assurée par les pompiers, volontaires ou professionnels.

pour affiner les derniers détails de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP). Ces quelques mois qui nous séparent de l’événement devront vous aider à parfaire votre plan de sécurisation. Pourtant, à cinq mois de la cérémonie d’ouverture, des interrogations demeurent. La France, à l’instar des sportifs, s’est elle suffisamment préparée ? Permettez moi de m’interroger, notamment s’agissant de la sécurité.

les Jeux ne sauraient se résumer à cette seule cérémonie, aussi grandiose soit elle. Les Jeux, ce sont deux semaines de compétition sur 39 sites répartis sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin, sans oublier les onze jours de compétition paralympique. Si la police et la gendarmerie sont rompues à la sécurisation des grands événements, avez vous l’assurance que les réservistes appelés en renfort le seront suffisamment ? Les nouveaux agents des entreprises de sécurité privées seront ils en nombre suffisant, alors que les difficultés de recrutement n’épargnent pas ce secteur ? été recrutés, avez vous l’assurance que la formation qui leur sera dispensée ne sera pas au rabais ? Par delà l’aspect sécuritaire, de la surveillance des organisations environnementales radicales, qui excellent dans l’art de s’appuyer sur des événements relayés en mondovision pour médiatiser leurs actions ? Enfin, comment comptez vous déjouer les cyberattaques, dont les conséquences seraient désastreuses si elles parvenaient à pénétrer nos réseaux en ligne ? Alors que l’olympisme rayonnera sur la France, nous n’avons pas le droit à l’erreur. À la moindre faille, notre prestige de puissance organisatrice s’évanouirait pour longtemps

De nombreux actifs dépendent des transports en commun pour leurs déplacements. Je pense précisément aux habitants de Seine Saint Denis, souvent des travailleurs de première ligne, qui prennent les transports pour de longs trajets. Si le Grand Paris Express, qui désenclavera notre département,

à l’afflux exceptionnel de voyageurs ? Quelles garanties le Gouvernement peut il apporter pour renforcer le réseau, en matière tant de signalétique que de gestion de flux ? Pouvez vous

Ma question portera sur la préparation de notre système de santé face à cet événement majeur. Un premier sujet est celui de la santé des athlètes, avec la polyclinique olympique et paralympique, gérée par Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP HP) et les hôpitaux de recours pour les athlètes et la famille olympique.

Nous savons tous qu’il y aura des risques majeurs, notamment en matière d’accueil, mais également de sécurité et de cybersécurité. Éviter la saturation de notre système de santé n’a rien d’aisé, quatre ans après le choc de l’épidémie de covid 19 et alors que l’été est normalement une période calme pour les hôpitaux. Comment comptez vous garantir une offre suffisante en matière de santé pour les résidents de la région d’Île de France comme des autres régions hôtes ? Quelles seront les capacités d’accueil effectives dans les hôpitaux durant les mois de juillet et août prochain ? Comment comptez vous assurer aux centaines de milliers de touristes qui se rendront en France un accès approprié à notre système de santé s’ils tombent malades ou s’ils ont besoin d’une intervention non programmée ? Quelle mobilisation prévoyez vous pour la médecine de ville ? Vous le voyez, les sujets sont nombreux, et leur poids est considérable. Mais peut être le point le plus important pour nous est la garantie des soins d’urgence, car nous savons tous que,

parer aux besoins de soins des différents athlètes, des accrédités, de la famille olympique, ainsi que des visiteurs – ils seront 12 millions pendant les jeux Olympiques sur notre territoire –, sans pour autant dégrader l’offre de soins pour les usagers habituels de notre service public hospitalier.

dans les différentes disciplines. Nous aurons également un réseau hospitalier composé de l’hôpital européen Georges Pompidou pour la famille olympique, de l’hôpital Avicenne pour les médias et de Bichat pour nos athlètes.

C’est important. Nous avons, en même temps, besoin d’affiner les besoins en urgentistes de la polyclinique. C’est le sens du travail que nous sommes en train d’achever avec le Comité d’organisation. Nous réfléchissons aussi, avec Frédéric Valletoux,

téléspectateurs, et nous attendons à peu près 15 millions de touristes sur les différents sites. Ces chiffres appellent une grande responsabilité à tous les niveaux, et l’image de la France, mes chers collègues, est manifestement en jeu. Madame la ministre, vous même

conformer à cette obligation légale. En ce qui concerne les hébergements, d’après les chiffres dont je dispose, moins de 3 000 chambres d’hôtel franciliennes sont officiellement accessibles. Le village olympique et les sites sportifs ont naturellement été conçus pour être accessibles, mais l’événement de taille que constituent les jeux Olympiques aurait pu être l’occasion d’accélérer

au métro, nous savons bien qu’il constitue le mode de transport le moins accessible à Paris. Il est important de contribuer à l’amélioration du réseau, en accord avec nos valeurs. L’accessibilité ne peut

pose également notamment M. Rémy Féraud, sénateur de Paris, et qui a trait à la société que nous voulons. Je veux parler de l’accueil et de l’hébergement des sans domicile fixe. Emmanuel Macron avait assuré, à l’été 2017, qu’il ne voulait plus personne à la rue d’ici à la fin de l’année. Les JOP doivent être l’occasion d’améliorer les conditions de vie des plus démunis. Quelles mesures avez vous envisagées pour cette population très particulière ? Monsieur le sénateur Kanner, je vous remercie de votre question, qui est vraiment l’occasion pour moi d’affirmer à quel point nous voulons que ces Jeux nous permettent de progresser dans l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, en pensant bien à tous les pans de l’expérience qui sera la leur, durant les jeux Olympiques comme pendant les jeux Paralympiques. Le recensement effectué par l’office de tourisme de la Ville de Paris à l’échelle de la métropole du Grand Paris, ce qui doit nous permettre de répondre à la demande en la matière. Nous avons prévu que 2 % des places soient spécifiquement réservées aux personnes en fauteuil roulant au cœur de nos sites, avec des des services dédiés qui leur permettront de se sentir bien et d’être bien accompagnées, en même temps que nous avons travaillé avec l’ensemble des préfets sur l’accessibilité des cheminements entre les gares. Je rappelle que 65 gares d’Île de France ont été rendues pleinement accessibles vers les sites de compétition.

Contrairement à ses voisins d’Europe du Nord, la France accuse un net retard dans la culture de l’accessibilité. Or, au moment où le monde entier aura les yeux braqués sur Paris et son organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la question de la place des personnes handicapées au cœur de cet événement sera primordiale. d’abord, l’accessibilité aux épreuves sportives, sommes nous prêts à accueillir les quelque 350 000 spectateurs en situation de handicap ? Je rappelle que, à l’intérieur de la petite couronne, seulement 9 % des stations du métro parisien leur seront accessibles ! Et, dans les bus équipés, seules deux places sont réservées aux voyageurs en fauteuil roulant…

Disposerons nous d’assez de « chambres PMR » pour les personnes en fauteuil roulant ? Selon les professionnels de l’hôtellerie, il n’y aurait que 3 500 chambres aménagées dans le Grand Paris, dont certaines seront sans doute utilisées par des pensionnaires valides… Le second point que je souhaite soulever est celui de la mobilité des personnes handicapées vivant dans les « zones rouges », interdites à la circulation automobile. Pour y circuler ou y être conduites, elles devront préalablement se déclarer en ligne. Étant donné que les plateformes de ce genre peuvent connaître des ratés lors de leur lancement et nécessitent d’être opérationnelles bien en amont, pouvez vous nous préciser la date de mise en service Enfin, si un habitant de la zone rouge est affecté, pendant la période des jeux, par un handicap, même temporaire, pourra t il s’inscrire rapidement sur cette plateforme ? La parole est à Mme la ministre. Je vous remercie de votre question, madame Ventalon. Je souhaite rappeler les différentes composantes de notre effort en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

dans nos infrastructures et dans nos sites sont réservées aux usagers en fauteuil roulant, qui feront l’objet d’une prise en charge spécifique par les équipes du Comité d’organisation.

voulons vraiment que les 65 gares qui ont été rendues accessibles en Île de France offrent un service plein, complet et satisfaisant aux personnes en situation de handicap.

dans nos sites, avec, encore une fois, des services spécifiques qui leur seront dédiés. Je tiens aussi à mentionner les efforts réalisés par les opérateurs en matière d’accessibilité universelle pour les déficients visuels et auditifs, avec des manchons en braille, et des braille, et des panneaux d’hypervision ou d’hypersignalisation, qui permettront un meilleur repérage. Je veux mentionner aussi la mise en place de la plateforme unique d’information et d’assistance en gare, prévue par la SNCF, ainsi que

Monsieur le sénateur Belin, je veux absolument m’inscrire dans la continuité de vos propos, pour saluer le travail mené par le Comité d’organisation, sous la houlette de Tony Estanguet, et vous dire

toutes les évolutions permettant que les transports soient à la hauteur. Je pense également à Michel Cadot et à l’ensemble de ses équipes, qui effectuent un travail considérable au service de la réussite des Jeux. Nous travaillons en équipe : une équipe de France,

Mme Christine Lavarde. Madame la ministre, dans un courrier daté du 30 janvier 2024 que le ministre Darmanin nous a adressé, il est écrit : « La sécurité constitue un défi que nous sommes capables de relever collectivement. […] Ce défi, c’est celui des agents du ministère. » J’ai envie d’ajouter : ce défi, c’est aussi celui des forces de police municipale, directement concernées, notamment dans les communes qui accueillent des sites olympiques ou en sont limitrophes

Mme la ministre.

confirmer que les crèches du ministère de l’intérieur et celles du ministère des armées seront disponibles. La Ville de Paris est également en train de finaliser une proposition en ce sens, pour nous permettre d’améliorer l’offre. Stanislas Guerini

Madame la ministre, le 5 janvier dernier, à l’appel de la chambre syndicale des buralistes d’Île de France, une opération coup de poing a été organisée, afin de dénoncer le fléau de la vente de cigarettes à la sauvette. Des cigarettes frelatées, imitées, sont vendues chaque jour un peu partout, provoquant leur lot de violences tout en posant un un véritable problème de santé publique. Ce trafic a explosé depuis quelques mois, au point de devenir un véritable phénomène de société, autant qu’un problème endémique de sécurité. Les buralistes, qui perdent du chiffre d’affaires, mais aussi de nombreux élus et riverains, qui connaissent des points de solidement installés dans leurs communes, le plus souvent à proximité des stations de métro ou des gares, créneau. La situation ne semble pas sous contrôle. Paris concentre une partie des points de vente illicites, avant les départements de Seine Saint Denis et du Val de Marne, mais le phénomène touche près de soixante dix départements selon la chambre syndicale des buralistes. Ce marché noir représenterait

illusoires. À l’approche des jeux Olympiques, la crainte est grande de voir ce trafic s’amplifier. Le préfet de police de Paris a certes annoncé un plan de lutte contre les ventes à la sauvette, mais la vente des cigarettes de contrebande est un problème en soi, qui se pose bien au delà de Paris intra muros. L’État doit enfin prendre très au sérieux ce phénomène national et y consacrer des moyens, en créant, par exemple, une brigade spécialisée dans les départements les plus atteints. Madame la ministre, je vous remercie de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous comptez prendre à différents échelons face à ce fléau.

n’y a pas besoin d’une disposition législative spécifique pour permettre à la fonction publique territoriale d’accorder des primes si les employeurs le souhaitent. Dans la fonction publique d’État, il n’y aura pas de prime JO. Nous n’avons pas besoin d’une assise spécifique ou d’une loi pour prévoir des primes. Nous nous appuyons sur les régimes indemnitaires existants. Chaque autorité employeuse est en mesure de procéder aux

je vous remercie

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un siècle après la toute dernière édition des jeux Olympiques d’été dans notre pays, nous aurons la chance d’accueillir, dans 143 jours précisément, le plus grand événement sportif et social de la planète.

Roland Garros, qui fait partie des plus grands et des plus prestigieux tournois de tennis du Grand Chelem, ou le Tour de France, qui est l’un des événements les plus regardés au monde. Nous sommes aussi régulièrement le pays hôte de compétitions internationales de football, de rugby et de championnats de ski alpin, etc.

Cojop, à commencer bien sûr par la livraison dans les temps et les budgets de tous les équipements olympiques et du village qui accueillera les athlètes et les médias. nous pouvons nous féliciter de la livraison par la Solideo de près de 68 ouvrages réalisés grâce à des entreprises françaises, lesquels nous permettent aujourd’hui d’avoir l’assurance que les compétitions pourront bien se dérouler dans de bonnes conditions. sont un défi logistique, mais ils se veulent également plus paritaires, écologiques, engagés, inclusifs, sobres et fédérateurs. De fait, même si certaines disciplines restent unisexes, il s’agira pour la première fois de Jeux totalement paritaires : 5 250 femmes et 5 250 hommes y participeront. Une attention particulière est portée aux émissions de carbone. Paris 2024 a, pour la première fois dans l’histoire des Jeux, fixé

La décentralisation de ces Jeux sur l’ensemble du territoire est une autre démarche remarquable, que je tiens à souligner. À cet égard, je salue la volonté du Cojop de faire de ces jeux non pas seulement les Jeux de Paris, mais ceux de toute la France. Je puis témoigner de l’engouement suscité dans notre département, en amont des jeux Olympiques, la possibilité d’accueillir des compétitions sportives et des centres de préparation et d’entraînement, ainsi que celle d’organiser des événements de promotion du sport, grâce au label Terre de Jeux, dont nombre de collectivités territoriales se sont emparées. Dans cet esprit de valorisation non pas seulement de Paris, mais de tout notre pays, le prochain temps fort est évidemment le relais de la flamme olympique, qui permettra de jeter la lumière, si je puis dire, sur l’histoire et le patrimoine français. Gageons que cet élan territorial se traduira par une promotion durable de la pratique du sport partout dans notre pays, où, comme ailleurs, l’obésité progresse à une allure préoccupante, particulièrement chez les jeunes. À ce sujet, madame la ministre, vous n’avez pas répondu aux craintes de Michel Savin concernant les coupes

attendu dans l’opinion publique. En effet, selon un récent sondage, seuls 59 % des Français ont l’intention de suivre cette Olympiade, alors même que près de 4 milliards de personnes à travers le monde Sans doute quelques problématiques évoquées cette après midi en séance ont elles contribué à cette réserve générale. En bref, il s’agit de la sécurisation de la cérémonie d’ouverture, évoquée notamment par notre collègue Catherine Dumas

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française, présentée par M. Pascal Allizard et plusieurs de ses collègues Dans la discussion générale, la parole est à M. Pascal Allizard, auteur de la proposition de loi. Monsieur le

de l’industrie de défense. Les amendements adoptés en commission visent à détailler et à préciser les contours du dispositif envisagé. Leurs dispositions lèvent à mon sens certaines incompréhensions nées chez les tenants du logement social et de l’environnement, au financement desquels, je l’indique d’ores et déjà, le présent dispositif ne portera pas atteinte. En ce qui concerne la raison d’être du dispositif, je rappelle que, après la supposée « fin de l’histoire » et l’époque de la « mondialisation heureuse », certains États – on peut le déplorer – réimposent des relations internationales fondées sur les seuls rapports de force, et non sur le droit, et s’appuient sur des narratifs nationalistes, voire belliqueux. Pour nous, les Européens, habitués aux dividendes de la paix, c’est la douche froide et le retour brutal aux réalités. Ces réalités, c’est le retour des tensions et de la guerre dans l’environnement proche de l’Europe largement démilitarisée.

En face, les Russes proposent ce qu’ils maîtrisent le mieux depuis longtemps : une guerre de saturation et d’attrition, appuyée par des moyens hybrides multiples. Notre voisin, le Royaume Uni, qui restait avec la France la seule puissance militaire en Europe, rencontre désormais les plus grandes difficultés avec les capacités de son armée et de ses industries. Quant aux Américains, ils pourraient revoir leur soutien à l’Europe après la présidentielle de 2024. Retrouver des forces morales, disposer de moyens financiers, humains et matériels significatifs, renforcer le lien entre l’armée et la Nation : tels sont les principes qui ont servi d’aiguillons à la préparation de la loi relative Madame la ministre, vous le savez, le Sénat a contribué de manière positive à l’élaboration de ce texte et il exerce un contrôle scrupuleux sur son exécution budgétaire. Or qui dit effort de guerre, économie de guerre et souveraineté dit aussi nécessité de disposer d’une industrie de défense performante et autonome. En matière de défense, la France peut s’enorgueillir d’avoir su conserver un modèle complet d’armée, mais également une base industrielle et technologique de défense (BITD) allant des grands groupes mondialisés aux PME locales, en passant par des start up, soit environ 4 000 entreprises. Cette BITD nous assure une capacité d’agir en toute indépendance, en cohérence avec nos ambitions stratégiques et notre modèle d’armée. Pourtant, plusieurs problèmes viennent assombrir l’avenir de ce secteur, l’un des derniers écosystèmes industriels français, indispensable à toute souveraineté et à la protection de la Nation. Ces dernières années, la question du financement des entreprises de l’industrie de Au départ, l’État était dans une certaine forme de déni : la défense ne représentait pas une priorité gouvernementale. Elle avait d’ailleurs parfois plutôt servi de variable d’ajustement dans les budgets du pays.

Des cas de refus explicites de financement ou d’ouverture de compte en raison d’une appartenance au secteur de la défense ont été signalés, et même des enregistrements produits, dans la mesure où ces refus sont parfois présentés oralement. Il n’existe aucune obligation pour les établissements bancaires de motiver leurs refus de financement. Certaines entreprises ne veulent pas communiquer sur le sujet, pour ne pas divulguer d’informations sur leur santé financière à de potentiels concurrents ou prédateurs. Des groupes bancaires ont fait le choix d’exclure purement et simplement les entreprises du secteur de la défense de leur politique d’investissement. D’autres excluent le soutien au commerce des « armes controversées

La Banque européenne d’investissement (BEI), institution publique, a également exclu de son champ de financement les munitions et les armes, ainsi que les équipements ou infrastructures militaires ou policiers, sans véritable base textuelle.

de ceux qui ne font pas partie de la chaîne de fournisseurs de ces grands groupes industriels. À la suite de la crise sanitaire, les grands groupes ont aussi pris conscience des risques pour la pérennité de leurs propres activités que représente la défaillance de leurs sous traitants et fournisseurs, en particulier les plus critiques, faute de financement. Ce fut notamment le cas de la filière aéronautique. Le contexte réglementaire complexe dans lequel les banques évoluent est régulièrement mis en avant pour justifier leurs réticences. il est vrai, faire face à deux risques principaux : un risque juridique, lié à l’application ou à la surinterprétation de règles environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et un risque réputationnel, entretenu par des lobbies qui incitent, souvent de manière agressive, à se désinvestir du secteur de la défense, sur le fondement de raisons prétendument éthiques. Nos banques d’envergure internationale sont les plus exposées. Le financement d’opérations d’export est particulièrement difficile pour des entreprises disposant pourtant d’une autorisation de l’État sous la forme d’une licence d’exportation délivrée, après une procédure rigoureuse, par la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels Ces travaux parlementaires ont permis d’objectiver le phénomène, d’appeler l’État à agir et d’inviter au dialogue entre deux mondes qui se connaissaient mal : d’une part, la finance, portée aujourd’hui par la finance verte, mais aussi, depuis toujours, par un besoin de retour sur investissement rapide ; d’autre part, l’industrie de défense, avec des spécificités qui peuvent inquiéter les banques, comme la dépendance à la commande publique, les cycles longs, les investissements souvent lourds, la rentabilité faible, les exportations vers des pays « exotiques

Puissance publique, banque, investisseurs privés, épargnants… Ne négligeons aucune piste ; il y va aussi de la résilience de la Nation

Je tiens d’ailleurs à saluer tout particulièrement Pascal Allizard, auteur de la proposition de loi, et Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui est également rapporteur pour avis. Tous les trois, nous avons travaillé ensemble pour enrichir le texte que nous examinons aujourd’hui. Je les remercie de leur implication. Ils alertent depuis de nombreuses années sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises de l’industrie de défense, pourtant cruciales pour notre sécurité, mais aussi pour notre économie. S’ils ont parfois eu l’impression que leurs alertes ne rencontraient que peu d’écho, les choses commencent, semble Quels sont les besoins de financement de ces entreprises ? J’en distinguerai trois. Le premier, c’est l’accès au crédit, le financement bancaire, essentiel pour la gestion par les entreprises de leur trésorerie, de leurs stocks et pour la modernisation de leurs chaînes de production. Sur ce point, les acteurs entendus en audition se sont accordés pour dire que les choses vont mieux depuis deux ans, le début de la guerre en Ukraine ayant marqué un vrai changement d’approche. Je relève ici l’apport du réseau des « référents défense » dans les grands établissements bancaires, en lien avec la Pour autant, aller mieux, ce n’est pas aller bien. Certaines entreprises font encore face à la frilosité des banques, qui craignent pour leur image ou imposent des exigences de conformité bien au delà de ce que prévoient les textes. Le deuxième enjeu, c’est l’accompagnement à l’export. Les contrats sont complexes. Là aussi, les banques sont parfois réticentes à se lancer dans ces dossiers. Plusieurs outils ont néanmoins été mis en place par la puissance publique pour accompagner les entreprises, par l’intermédiaire de garanties et d’assurances. Ces dispositifs sont gérés au nom et pour le compte de l’État par Bpifrance Assurance Export. S’ils sont ouverts à l’ensemble des sociétés, ils bénéficient plus particulièrement aux entreprises de la défense. Le secteur militaire représente 40 % des encours de crédits export garantis, qui s’élevaient à 65 milliards d’euros en 2022. Le troisième enjeu, et le plus pressant aujourd’hui, ce sont les fonds propres. Cette difficulté est loin d’être réglée. Elle affecte de manière disproportionnée les entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Le capital investissement est quasiment inexistant dans le secteur de la défense en France et en Europe. Les outils publics gérés par Bpifrance se révèlent insuffisants pour combler les faiblesses du secteur privé. Or, faute d’un volume d’investissements suffisant, les entreprises de la BITD n’ont pas d’autre choix que de renoncer à leurs projets ou de se tourner vers des financements extraeuropéens.

Ensuite, le signal envoyé par les institutions européennes est particulièrement négatif. Le Fonds européen d’investissement (FEI) de la BEI interdit de financer les munitions, les armes, ainsi que les équipements ou infrastructures militaires ou policiers. Surtout, il impose ces exclusions aux fonds d’investissement qui participent à ses tours de table. Par ailleurs, même si la France a obtenu la mise en place d’un mécanisme de fonds propres dans le domaine de la défense, celui ci est réservé aux seules entreprises dont moins de 50 % du chiffre d’affaires sont liés à la défense. Cette attitude, mes chers collègues, est d’autant plus inexplicable – j’insiste sur ce point – que le commissaire européen Thierry Breton parle de consacrer 100 milliards d’euros à la défense et que la présidente de la commission, Mme von der Leyen, affirmait récemment que l’enjeu des prochaines années pour l’Europe était la défense. Enfin, la France se heurte aux réticences de certains de ses partenaires européens ; je pense notamment à l’Allemagne. J’espère néanmoins, et Mme la ministre pourra nous le confirmer, que la France continuera son action pour assouplir la doctrine d’intervention de la La proposition de loi s’inscrit dans ce contexte et entend apporter une première réponse aux difficultés de financement. Elle prévoit de flécher une partie des encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) non centralisés auprès de la Caisse des dépôts vers le financement des entreprises

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Sénat est amené à examiner ces deux dispositions. Elles ont été votées à deux reprises par notre assemblée, en loi de programmation militaire et en loi de finances pour 2024. C’est grâce à la commission des affaires étrangères et de la défense que le sujet avait été avait été introduit dans la LPM. Or, dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a censuré les mesures adoptées, pour de strictes raisons de forme, considérant qu’il s’agissait de cavaliers. Cette difficulté est désormais levée, avec un véhicule législatif propre.

dans le projet de loi de finances pour 2024, pour lequel il avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 je terminerai en vous présentant les trois grandes modifications apportées par la commission au texte initial de la proposition de loi. Tout d’abord, nous avons réécrit l’article 1, afin que le nouvel objectif de financement des entreprises de défense n’empiète pas sur les cibles aujourd’hui allouées aux encours non centralisés du livret A et du LDDS. Je sais que cela répondra à l’inquiétude de plusieurs d’entre vous : les sommes allouées au financement de la transition écologique et de l’économie sociale et solidaire ne sont en aucun cas concernées. nous avons explicité les missions de Bpifrance en faveur des entreprises de l’industrie de défense française. Opérateur du soutien au financement des entreprises et de l’innovation, Bpifrance gère aujourd’hui de très nombreux dispositifs de soutien aux entreprises. Pour autant, depuis sa création, en 2005, le contexte géopolitique a évolué. Il nous paraît important de mentionner sa contribution à l’économie de guerre, dans le droit fil de la LPM. Enfin, nous avons complété le rapport prévu à l’article 2 de la proposition de loi. Cette évaluation est primordiale. Elle doit permettre tant d’avoir une idée objective des besoins de financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense que d’aborder l’ensemble des problématiques auxquelles ces entreprises peuvent être confrontées. Le rapport sera l’occasion de passer en revue les outils existants et d’évaluer l’opportunité d’en créer de nouveaux. Je pense ici, par exemple, aux garanties et assurances à l’export, à des outils de renforcement des fonds propres ou encore à la création d’un plan d’épargne dédié au secteur de la défense, qui fait d’ailleurs l’objet amendements. Il est nécessaire de disposer au plus tôt des outils les plus appropriés. Enfin, au regard de l’importance de la réglementation européenne sur les critères ESG et de son impact sur les entreprises de la défense, le Gouvernement devra présenter les actions qu’il a menées pour que le financement de la défense soit davantage pris en compte, y compris au sein de la Banque d’investissement. Mes chers collègues, je vous appelle désormais à soutenir ce texte, qui envoie un signal politique clair aux acteurs financiers et institutionnels en faveur du soutien aux entreprises de notre industrie de défense. La parole

est forcément favorable. Depuis 2020, notre commission a alerté, en particulier par la voix de Pascal Allizard, auteur de cette proposition de loi, sur les difficultés de financement de notre industrie de défense. Nous avions proposé dans la loi de programmation militaire de créer un nouveau livret d’épargne. Réécrit en commission mixte paritaire, le dispositif avait pris la forme d’un fléchage d’une partie des encours de l’épargne réglementée. Réintroduit par un amendement de nos collègues députés dans le dernier projet de loi de finances, il avait même été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité. Si nous en rediscutons aujourd’hui, ce n’est donc pas du fait d’un désaccord entre les assemblées ou entre le Parlement et le Gouvernement. C’est parce que le Conseil constitutionnel a considéré que ce dispositif n’avait sa place ni en LPM ni en loi de finances. L’analyse selon laquelle le dispositif de financement des entreprises de la défense n’avait aucun lien, même indirect, avec le chapitre de la LPM consacré à « l’économie de guerre » laisse songeur. Mais telle a été la décision Revenons en au fond. Quel est au juste le problème de financement de notre BITD ? Il comporte deux volets. Le déficit de fonds propres est le mieux documenté. En un mot, l’écosystème de financement est faible, car les investisseurs connaissent mal le secteur et craignent de s’y intéresser. Mais nos entreprises, surtout les plus petites d’entre elles, rencontrent aussi des difficultés d’accès au crédit. Parce que le problème n’est pas facile à mesurer, il est nié, à la fois par le secteur bancaire, par la direction générale du Trésor et par la Banque de France. Mais la difficulté n’en est pas moins réelle. La « frilosité bancaire » à l’égard de la défense est attestée depuis 2020 par la DGA, par les industriels eux mêmes, par au moins deux rapports de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dernièrement, par la Cour des comptes. Comment y remédier ? Soit par un produit s’apparentant à l’épargne réglementée, c’est à dire liquide et connue pour cela des Français. Ce serait un moyen commode de financer les besoins de court terme des entreprises. Soit par un produit spécifique soutenant l’investissement en fonds propres par l’acquisition de titres. Cela répondrait à un problème mieux identifié, mais par un placement moins liquide et plus risqué, donc destiné à un public d’épargnants plus choisi et désireux de financer ce secteur. La première solution, celle du livret A, a déjà été validée deux fois par le Parlement, dans la LPM et dans le PLF. C’est la plus à même de s’attaquer au problème commun à toutes les difficultés de financement, c’est à dire à la conformité excessive du monde financier aux critères d’investissement responsable, les fameux critères ESG. Comme l’a souligné en commission le rapporteur Dominique de Legge, dont je salue le travail et que je remercie de son écoute attentive et de son implication pour trouver des solutions efficientes, aucune norme, aucune taxonomie, aucun écolabel ne mentionne la défense. C’est donc largement du fait d’un halo négatif entourant le secteur que le monde financier rechigne à y investir ou que telle caisse régionale refuse, par crainte pour sa réputation, d’ouvrir un compte à une start up. Disons le très clairement : dans un contexte géopolitique qui ne cesse de se dégrader, cet implicite négatif sape l’effort de redressement de notre outil de défense Faire de la BITD une priorité dans l’allocation de l’épargne préférée des Français serait un signal fort à l’attention des acteurs de la finance. au problème de l’apport en fonds propres, il faut structurer le secteur et faire évoluer la doctrine de la BEI, afin d’entraîner la communauté des investisseurs. Le texte a parfois suscité des craintes infondées. Tout d’abord, la menace pesant sur le financement du logement social est tout simplement inexistante, puisque les encours visés sont ceux qui ne sont pas centralisés à cette fin à la Caisse des dépôts. autre risque parfois invoqué est celui de la décollecte, au motif que les épargnants pourraient être réticents à financer la production d’armes. Eh bien oui ! Nous en avons déjà parlé lors de l’examen de la LPM : rien ne permet d’étayer cette crainte,… Ah bon ? … et l’objet du texte est précisément de banaliser l’idée même d’investir dans la défense. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas laisser la bancaire empêcher davantage notre industrie de la défense de se développer. L’heure est grave. On nous parle d’économie de guerre, de 200 000 emplois directs, de 4 000 PME et ETI sur le territoire national dans nos territoires. Aussi, donnons à notre BITD les moyens de se développer. Faisons de notre défense et de notre sécurité notre priorité ! La commission des affaires étrangères et de la défense soutient donc fermement cette initiative. La

cette proposition de loi s’adresse aux entreprises de l’industrie de la défense française et cherche à améliorer leur financement au travers du fléchage d’une partie des ressources collectées au titre du livret A

Le Gouvernement est très attentif aux besoins de financement du secteur de la défense. Ils sont importants et croissants. Depuis 2020, plusieurs rapports parlementaires

Face à ces alertes, le Gouvernement a mobilisé les services de l’État pour identifier les freins au financement du secteur. En septembre dernier, des « référents défense » ont été mis en place pour mettre en contact, le ministère des armées, des banques françaises avec les entreprises de la BITD rencontrant des difficultés pour obtenir un crédit. Un travail en profondeur a également été mené par la direction générale du Trésor auprès des industriels comme des banques, pour établir un diagnostic des freins existants. Les conclusions de ces travaux sont, me semble t il, assez éclairantes. Les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la BITD pour obtenir un crédit bancaire ne sont, dans la plupart des cas, pas liées au fait que l’entreprise appartienne au secteur de la défense. Certaines ont rencontré des difficultés pour obtenir un crédit. Mais, d’après les études dont nous disposons et le travail en profondeur de la direction générale du Trésor, c’est majoritairement pour des raisons économiques, économiques, et non par discrimination du fait de leur appartenance au secteur de la défense. En revanche, il apparaît très clairement que les difficultés sont bien plus importantes pour les PME de la BITD quand il s’agit d’accéder au financement

les banques – certes, il y a toujours des exceptions – suivent majoritairement les PME qui ont des projets, mais les capitaux, eux, ne sont pas aussi facilement disponibles, voire sont indisponibles.

que les matériels de guerre soumis au contrôle à l’export ne soient pas soumis aux dispositions de la directive sur le devoir de vigilance. Face à de tels constats, le fléchage de l’épargne réglementée ne nous semble pas être la solution adaptée pour améliorer le financement de l’industrie de défense. d’abord, parce que flécher les emplois du livret A et du LDDS vers la BITD ne résoudrait pas nécessairement le problème d’accès à des financements en fonds propres, étant donné que les obligations d’emplois concernent des prêts et que, vous le savez, les dépôts des Français, disponibles à tout moment, ne peuvent être immobilisés dans des investissements en fonds propres. Ensuite, permettez moi de rappeler à votre sagacité que le bilan des banques est fongible. L’ensemble des ressources des banques financent l’ensemble des emplois, et ces établissements ne sont pas en mesure d’affecter directement un dépôt à des usages spécifiques. Compte tenu du fait que l’industrie de défense est un petit secteur très spécifique, flécher une partie de l’encours de l’épargne réglementée vers elle ne répondrait pas aux besoins de dispositifs sur mesure. Néanmoins, soyons clairs : ainsi que vous l’avez compris, le Gouvernement accueille favorablement la volonté du Sénat d’envoyer le signal fort sur les besoins de financement des PME de la défense. De ce point de vue, nous sommes favorables au principe d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le diagnostic, sur les solutions envisagées au niveau national

dans le cadre du débat parlementaire. Sur le fond, le Gouvernement souhaite poursuivre les efforts pour améliorer l’accès aux financements en fonds propres, qui sont lacunaires. Le ministre de l’économie entend tout d’abord réunir à l’été, en lien avec le ministre des armées, les acteurs financiers, mais aussi les investisseurs et les industriels de la défense, pour un événement majeur sur le financement du secteur de la défense et l’augmentation des fonds propres de nos PME. L’objectif sera de lever les préventions des gestionnaires de fonds, mais aussi de lancer un forum permanent entre acteurs financiers de la place et industriels de la défense. Nous pensons que la Caisse des dépôts et consignations, mais également Bpifrance, aura un rôle particulier à jouer en la matière. Par ailleurs, nous poursuivrons nous poursuivrons l’action entreprise depuis 2017 à la BEI, pour qu’elle finance plus fortement l’effort de souveraineté européen, qui a déjà pris de l’ampleur sur les projets avec composante duale. Il convient de saluer le lancement en janvier 2024 par le FEI, bras armé en capital de la BEI, d’un mécanisme de fonds propres dans le domaine de la défense, doté de 175 millions d’euros, même s’il conserve clairement des limitations très, voire trop importantes. Pour que le groupe BEI fasse davantage dans ce secteur, il faudra faire évoluer sa politique de prêts.

donne l’occasion de porter la modification de la liste d’exclusion et de l’assouplissement des critères d’éligibilité des entreprises. Bruno Le Maire, qui est le gouverneur français pour la BEI, a bien cet élément en tête. Enfin, le Gouvernement entend aussi mener une revue des dispositifs publics qui soutiennent l’accès aux fonds propres de nos PME et ETI de la défense. Là où il sera nécessaire et utile de les renforcer, nous proposerons de le faire, afin de catalyser plus d’investisseurs privés vers ce secteur primordial. Sur tous ces travaux,

de cavalier législatif n’est pas anodine : c’est le symptôme d’une volonté de passer en douce, par effraction, pour faire main basse sur l’épargne populaire des Français. Oui, nous assistons aujourd’hui à une tentative de flibusterie sur l’épargne réglementée. Vous souhaitez utiliser les encours non centralisés du livret A et du livret de développement durable et solidaire pour financer la BITD. Pour le dire simplement : financer les marchands de canons en prenant dans les livrets avec lesquels les Français pensaient financer le logement ou le développement durable

Notons que l’État a des participations dans la BITD, l’agence des participations de l’État – cela représente tout de même 30 % de son portefeuille –, et que Bpifrance et la Caisse des dépôts ont également déjà des participations dans le secteur. Notons également qu’il existe de nombreux fonds d’investissement publics ou privés et que l’État a mis en place

la création de l’AID, avec son guichet destiné à structurer la filière innovation défense. Le résultat ? Une grande dynamique des commandes à l’export : 27 milliards d’euros en 2022, un chiffre inégalé ! Plus structurellement, le secteur de la défense a connu les mêmes évolutions que le reste de la sphère privée du pays financiarisation, recherche accrue du profit. La différence majeure avec les autres activités – chacun pourra le constater – est que le secteur reste biberonné de manière intense par la commande publique, notamment la direction générale de l’armement. Alors oui,

mes chers collègues, s’il y a un problème à ce sujet, c’est parce que l’investissement privé fait défaut. Ce sont les banques qui sont frileuses, principalement parce que l’industrie de défense n’est pas une activité qui entre dans les critères ESG. C’est donc avant tout un problème d’image et d’éthique, qui doit se régler avec les banques. Pourquoi, si même les banques et les investisseurs privés sont réticents, serait ce à l’épargne réglementée des Français de combler les trous ? On a beaucoup parlé aussi des technologies duales, pour souligner les bénéfices apportés par le secteur de la défense. Mais si, dans les années 1950, la défense était le leader de l’innovation, avec 60 % du total des technologies portées à maturité du pays,

Rappelons que le livret d’épargne a été créé en 1818 pour reconstruire le pays après les ravages causés par les guerres napoléoniennes. Oui, le boucher de l’Europe à l’époque était français ! On est donc dans un esprit diamétralement inverse à celui de la proposition aujourd’hui : il s’agit historiquement d’un outil financier créé par et pour la paix. L’objectif principal du livret A, connu de tous, celui pour lequel ce produit reste populaire, c’est de financer le logement social. S’il faut réformer faut le faire vers l’augmentation de la recentralisation des encours pour soutenir ce secteur, au vu de la crise du logement que traverse le pays. S’il y a une ouverture sur les encours, nous estimons bien plus urgent de flécher ceux ci vers le logement plutôt que vers les marchands de canons. Enfin,

peu confuses. Parmi vos arguments figure en effet le conflit en Ukraine. Si l’enjeu est de soutenir l’effort de guerre ukrainien, alors il faut le dire et instaurer une clause de revoyure au regard de la situation sur place. Nous en sommes convaincus : l’épargne réglementée des Français doit avoir

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dès le 13 juillet 2022, le Président de la République Emmanuel Macron utilisait l’expression d’« économie de guerre

Le projet guerrier sous tendu par la marchandisation et la spéculation sur les ventes d’armes a fait de notre pays le troisième exportateur d’armes au monde, pour un montant de 49,9 milliards d’euros entre 2000 et 2022. Nous proposons de réduire la part du chiffre d’affaires à l’export de nos entreprises de défense à 30 %. La souveraineté ne se décrète pas ; elle se construit sur un projet politique cohérent. en place d’un pôle public de l’armement, en renforçant les prises de participation dans des TPE PME de la base industrielle et technologique de défense. Cela doit d’abord se faire le bras financier de l’État,

sur les 24 milliards d’euros d’achats du ministère des armées, seuls 11,74 milliards d’euros de commandes publiques aient bénéficié à notre industrie. Pire, les microentreprises et les PME industrielles n’ont capté que 538 millions La sous traitance en cascade dilue les responsabilités et prive les TPE PME de la valeur ajoutée ; c’est également vrai dans le secteur de la défense. Quoi de mieux que de produire et de vendre pour financer ses investissements ? L’argument de la frilosité des banques n’a par ailleurs jamais été démontré. Il ne l’a

Il est préférable d’en rester à ce que l’épargne réglementée, qui est en France et de très loin la plus développée d’Europe, réalise bien ». En responsabilité, notre groupe votera contre cette proposition de loi, qui nous semble inappropriée et dangereuse.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après bien des péripéties, nous voilà réunis aujourd’hui pour débattre du financement des entreprises de défense de l’industrie française.

ma position, avec comme ligne de conduite la seule promotion d’un lien fort entre la Nation et ses armées.

Or ce contexte a fortement évolué : avec l’invasion de l’Ukraine, la guerre est revenue aux portes de l’Union européenne. Nous pouvons le déplorer ou feindre de l’ignorer, mais c’est une tragique réalité. Regretter que la paix par le droit ne soit plus qu’un vœu pieux, en soupesant nos aveuglements depuis la fin de la guerre froide, ne doit pas nous réduire à la procrastination. Un relatif consensus s’était établi pour constater que notre outil de défense, comme dans bon nombre d’États, était adapté à des temps de paix et de politiques interétatiques laissant place au dialogue et à la diplomatie. En revanche, entrer dans une économie de guerre suppose, pour les entreprises de la BITD, et en particulier les PME, de disposer des fonds nécessaires, en complément d’un effort budgétaire réel, favorisé par d’importants investissements. Si l’agression russe a réveillé l’Europe stratégique, la menace doit bousculer notre naïveté, aussi légendaire que nos inerties coupables. Plus que des paroles ou des discours, des financements pérennes rendront crédibles nos positions de fermeté. C’est pourquoi j’assume la responsabilité de cosigner cette proposition de loi, ainsi que

Ensuite, nul ne conteste que les entreprises de la défense, principalement les PME, connaissent des difficultés d’accès au crédit. Ces freins sont liés liés à la question de l’éthique de la fabrication des armes, laquelle serait, comme l’écrit si bien Pierre Louis Boyer, « le piège contemporain de l’efficience morale ». Cette vision morale peut se comprendre. Est elle cependant acceptable et soutenable face à la montée des périls ? Voilà plusieurs décennies, François Mitterrand regrettait que les missiles soient à l’est et les pacifistes à l’ouest. Devrons nous nous contenter d’être des professeurs de morale ?

Avec ce texte, nous offrons la possibilité aux épargnants français de donner sens à ce combat pour défendre nos valeurs et nos idéaux, malmenés et menacés par le cynisme et la force brutale de dirigeants dérangés et sans scrupules. Ils savent mieux que quiconque que l’argent est le nerf de la guerre. En ouvrant ces ces possibilités de financement, nous ne laissons pas nos sentiments bellicistes l’emporter. Nous faisons simplement preuve, mes chers collègues, de cohérence. En ces temps incertains,

Reconnues notamment pour leur qualité, ces pépites technologiques françaises suscitent déjà un fort intérêt chez les investisseurs étrangers. Certaines d’entre elles rencontrent toutefois des difficultés de financement qui entravent leur développement, malgré l’intervention de l’État pour assurer leur sécurité financière, des contrats avec

souveraineté ». Les versements sur ce nouveau livret d’épargne réglementé devaient être affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie française, notamment des entreprises Bien que de petite taille en comparaison d’autres secteurs industriels, les industries de défense françaises concentrent néanmoins un savoir faire et un faire savoir uniques, dont notre pays tire une grande partie de sa puissance militaire. Cette filière d’excellence, non délocalisable, assure à la France une parfaite maîtrise de nombreuses technologies de pointe et se révèle cruciale pour garantir notre dissuasion nucléaire. Voilà quelques mois, la chambre haute approuvait la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, non sans alerter sur la nécessité de soutenir les entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Le ministre des armées, M. Sébastien Lecornu, avait notamment parlé de la nécessité de donner de la visibilité à notre BITD, de la protéger et de la promouvoir. Il avait également exprimé son soutien aux dispositions proposées par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat pour développer des mécanismes visant à mieux financer ces entreprises, en particulier les PME. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans ce contexte : elle prévoit, à l’article 1, de flécher une partie des encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire.

Les industriels ont souligné le rôle majeur joué par le réseau des référents défense au sein des grandes banques, en lien avec la DGA. Dans le même temps, certaines banques ont assoupli leur doctrine d’intervention dans le secteur de la défense. Plusieurs outils ont été mis en place par la puissance publique pour accompagner les entreprises, par l’intermédiaire de garanties et d’assurances. Ces dispositifs sont gérés, au nom et pour le compte de l’État, par Bpifrance Assurance Export. S’ils sont ouverts à l’ensemble des entreprises, ils bénéficient plus particulièrement à celles de la défense. Plus que jamais, la menace protéiforme internationale nous renforce, si cela était encore nécessaire, qu’il faut soutenir concrètement notre industrie de défense. Ce message n’a pas été seulement entendu par le Gouvernement. Il a heureusement été anticipé dès 2017, puisque nous aurons, au terme des deux mandats du Président de la République, plus que doublé le budget de la défense française. L’industrie française de défense est bien placée pour contribuer au réarmement et au renforcement de la souveraineté européenne. Il est impératif de bien prendre conscience et de faire comprendre qu’une BITD forte assure à nos armées, en toute indépendance, la capacité de défendre nos intérêts partout où la France se doit d’intervenir. se doit d’intervenir. Mes chers collègues, la France et l’Union européenne ont plus que jamais besoin d’une industrie de défense forte et performante. L’orateur Cicéron disait en son temps : « Quand les armes parlent, les lois se taisent.

et solidaire afin de soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur de la défense. Cette proposition soulève des enjeux majeurs qui touchent à la fois à nos priorités nationales et à nos valeurs démocratiques. Dans un monde multipolaire marqué par des tensions géopolitiques permanentes, la France, comme l’ensemble de ses voisins, se trouve confrontée à des défis sécuritaires de taille. La guerre est de retour, en Europe comme au Moyen Orient, et menace la souveraineté des nations. Ces troubles Ces troubles ont mis en lumière la nécessité impérieuse, pour notre pays, de renforcer ses capacités de défense. Dans ce contexte, il est regrettable que notre industrie ne soit pas en mesure de répondre à la demande croissante d’équipements militaires. En dépit des nombreuses revendications quant à la supériorité de notre armée en Europe, notre effort de défense restera limité à 1,9 % du PIB en 2024, soit moins que l’objectif établi par l’Otan. Je tiens à rappeler qu’en comparaison avec les pays européens, la France a réduit au minimum, ces dernières années, sa capacité à réagir souverainement aux conflits internationaux. Si la fin des dividendes de la paix nous presse d’agir pour garantir la sécurité de notre pays, elle ne doit pas faire oublier que cette situation est le résultat de choix politiques antérieurs. Malgré la nécessité de ce réarmement, je m’interroge sur la pertinence du véhicule retenu pour le financer, tant ce dernier soulève des préoccupations légitimes.

Le passage en économie de guerre, comme le revendiquent les auteurs de ce texte, est confiné au rang de mots dont on peine à comprendre les tenants et aboutissants concrets. Une telle mobilisation économique doit revêtir une certaine onction démocratique, tant elle redéfinirait les priorités nationales pour les mois et les années à venir. Or notre pays vit une crise du logement qui ne cesse de s’aggraver : on dénombre aujourd’hui près de 4 millions de personnes mal logées et 330 000 personnes sans domicile.

ce que nous dit la Fédération bancaire française, quand elle déclare que l’industrie de l’armement ne fait pas l’objet d’une stigmatisation particulière de la part des banques, mais que ses difficultés tiennent plus à la nature même des normes imposées au financement des activités de ces entreprises. On peine à comprendre en quoi agir sur le volume et le flux changera quoi que ce soit. Enfin, je tiens à rappeler que les investissements des Français en faveur du secteur de la défense sont d’ores et déjà en hausse.

Ce dispositif plus volontariste est nettement plus démocratique. Les entreprises du secteur de la défense, souvent victimes de la frilosité des banques à les financer, seraient aussi bien plus aptes à lever des fonds. Face à un sujet aussi sensible, notre conviction profonde est celle de la nécessité d’une approche équilibrée, réaliste, et respectueuse de nos principes fondateurs.

étant, si l’épargne des Français est l’une des plus importantes du monde, sa mobilité et sa performance posent question. Nos compatriotes plébiscitent majoritairement les placements prudents : épargne réglementée ou fonds en euros S’il ne nous appartient pas, en tant que législateurs, de changer les comportements de nos compatriotes, nous pouvons néanmoins agir sur la mobilité de ce capital. Au delà de l’aspect Au delà de l’aspect purement financier, l’épargne française est un atout qui peut et doit être mis au service de notre souveraineté. Certains grands gestionnaires d’actifs ne s’y trompent d’ailleurs pas en convoitant une manne financière qu’il leur tarde de faire vivre ailleurs. Citons aussi ces pays qui ont constitué des fonds souverains, aujourd’hui opérationnels et offensifs : Russie, Chine, Arabie saoudite, Qatar et Norvège. Ces structures sont devenues de véritables instruments de puissance dont leur État d’origine n’hésite pas à faire usage. Face à ces enjeux mondiaux, les pouvoirs publics, et plus particulièrement le législateur, doivent s’emparer du sujet. Nous devons faire de cette spécificité française un atout au service de nos petites et moyennes entreprises de l’industrie de défense.

Avec d’insuffisantes ressources propres, nos petites et moyennes entreprises de la défense sont plus que jamais exposées à des menaces de rachats hostiles ou de prises de participation étrangères, comme cela a été rappelé. Je pense par exemple à la pépite française Photonis, qui a longtemps été sous la menace d’un rachat par un groupe américain. Certes, le dispositif de contrôle des investissements étrangers assure un tamis protecteur, mais il n’est pas automatique et a déjà été pris en défaut par le passé. Très souvent, le blocage de Bercy pour les petites et moyennes entreprises est la conséquence indirecte de difficultés à croître au même rythme que la concurrence étrangère.

Depuis plusieurs décennies, la France a choisi une voie étroite, mais courageuse : celle de l’indépendance. Le prix à payer est de soutenir coûte que coûte notre BITD, afin de conserver les moyens d’une armée aux équipements et aux armements modernes. Si cela venait à faillir, nous serions obligés de faire comme nombre de nos voisins européens : acheter à l’étranger, au prix d’une perte d’indépendance et d’autonomie stratégique. Ainsi se profile l’équation à laquelle nous devons sans cesse trouver de nouveaux moyens de répondre. La présente proposition de loi devrait y contribuer et, à ce titre, je me réjouis de l’initiative de notre collègue Pascal Allizard. En Européenne convaincue mais vigilante, je souhaiterais également élargir le spectre de la réflexion. Avec le retour de la guerre à ses frontières, l’Union européenne avance ses arguments pour remettre en état une défense européenne. Plusieurs dispositifs ont été lancés par la Commission en ce les montants affectés s’envolent. L’ (Edirpa), par exemple, est déjà doté de 300 millions d’euros. De récentes déclarations font état, par ailleurs, d’une montée en gamme, à hauteur de 100 milliards d’euros, de la défense européenne. En complément du texte que nous examinons, c’est un soutien dont notre tissu de petites et moyennes entreprises pourrait profiter.

Saluons la volonté, mais restons prudents et fidèles à notre stratégie d’indépendance. Soyons pragmatiques et faisons bon usage également de nos différents instruments. En un mot, votons sans ambiguïté cette proposition de loi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà une semaine, le Président de la République déclarait que l’envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien ne pouvait être exclu. Depuis, exégèses et polémiques se multiplient, en France et même au delà de nos frontières. Force est de constater que l’exécutif a atteint son objectif : l’ambiguïté stratégique bat son plein. Une telle ambiguïté peut être lourde de conséquences, bien sûr, mais n’oublions pas que c’est Poutine, et lui seul, qui est le responsable de la guerre d’agression en Ukraine. Une chose est sûre pour entretenir cette ambiguïté stratégique, mieux vaut avoir de solides arguments, des arguments suffisamment robustes pour faire douter les puissances, qui, à défaut d’être nos ennemis directs, sont les ennemis de nos alliés. C’est pourquoi nous sommes très nombreux, ici, à soutenir le réarmement du pays. Nous l’avons récemment exprimé de façon univoque en votant, très largement, la loi de programmation militaire présentée par le Gouvernement. Avec plus de 400 milliards d’euros de dépenses prévues pour la période 2024 2030, l’effort est sans précédent. Je tiens, au nom du groupe Les Indépendants, de nouveau Le contexte international nous oblige à cet effort. Alors qu’une nouvelle aide des États Unis est bloquée par leur Congrès, les Européens prennent conscience du fait qu’ils pourraient bientôt être les seuls à soutenir, matériellement et moralement, l’Ukraine. En ce jour de outre Atlantique, Trump est en passe d’être désigné candidat officiel des Républicains pour la présidentielle de novembre prochain, et il a déjà recommencé à faire de la géopolitique à coups de expéditifs annonçant notamment la fin du soutien américain à l’Europe face à la Russie. Les Européens se rappellent désormais que, pour maîtriser leur destin, il faut que leurs nations se réarment. À cet égard, il est urgent de marquer le coup. Nous devons entrer en économie de guerre : la puissance publique doit intervenir dans le secteur économique pour indiquer les priorités stratégiques nécessaires au réarmement de la Nation. Notre commissaire européen, Thierry Breton, a déjà recouru à cette expression, dont il connaît parfaitement la portée.

Ce rapport, parmi nombre de propositions d’action très concrètes, recommandait, notamment, de mobiliser l’épargne privée pour massifier les financements de l’industrie de la défense. Depuis, l’idée a fait son chemin, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Elle a même été retenue par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2024.

C’est pourquoi je me réjouis que nous examinions enfin un véhicule législatif, ce qui devrait permettre d’éviter que la mesure ne connaisse encore le même sort. La mobilisation de l’épargne des Français doit devenir un outil de politique publique en phase avec nos objectifs stratégiques. C’est ce que le groupe Les Indépendants a déjà défendu à plusieurs reprises, et encore récemment avec l’adoption de ma proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises. est encore plus vrai depuis la crise sanitaire, la « surépargne covid » n’ayant pas disparu. Aujourd’hui, je le rappelle, les encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire avoisinent les 550 milliards d’euros. Au vu de notre endettement public, cette manne privée est considérable. À titre personnel, il me semble que la création d’un livret spécifique dédié au financement des entreprises de la défense aurait le mérite de la clarté et de la transparence pour les épargnants citoyens. C’est la ligne que notre groupe avait défendue dans ses différentes propositions qui prévoyaient de mobiliser l’épargne privée vers d’autres objectifs. Cependant, compte tenu de l’urgence de la situation, il me semble que la solution la plus efficace à court terme doit être privilégiée. C’est pourquoi la mobilisation d’une partie de l’enveloppe d’ores et déjà prévue pour le financement des entreprises nous paraît être, à ce stade, la mesure la plus pertinente. Notre groupe accueille donc très favorablement cette proposition de loi. Je vous présenterai tout à l’heure deux amendements qui s’inscrivent dans la même logique et qui visent à accélérer le passage à une véritable économie de guerre. La parole est à M. Michel Canévet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, est venu dire au Sénat combien l’Europe soutenait l’accroissement de l’effort des industries de défense

chers collègues,

Alors que les industries de défense françaises représentent plus de 4 000 entreprises et totalisent un chiffre d’affaires de près de 30 milliards d’euros, notre BITD fait face à des difficultés de financement qui pourraient entraver, à la fois, son développement et son avenir. Ces entreprises – grands groupes, start up ou PME – représentent plus de 200 000 emplois de haute technicité, non délocalisables. Elles participent également au dynamisme économique de nos territoires et permettent d’y maintenir compétences et emplois. La France a fait le choix, malgré de nombreuses contraintes budgétaires, de préserver et de renforcer un modèle d’armées complet, choix qu’elle a réaffirmé lors de l’élaboration et de l’examen de la dernière loi de programmation militaire. Une filière industrielle résiliente est donc nécessaire pour soutenir ce modèle. Même si le soutien de l’État et son rôle historique restent centraux, les difficultés s’accumulent : l’accès aux prêts bancaires demeure difficile et les fonds d’investissement dédiés à la défense sont trop peu nombreux. Ainsi, la capacité à obtenir des financements adaptés aux besoins est aujourd’hui au cœur des inquiétudes relayées par les armées et les industriels. Par ailleurs, la concurrence mondiale se durcit, avec des entreprises extracommunautaires souvent très soutenues par leurs États. Les entreprises françaises de l’armement suscitent de plus un fort intérêt de la part d’investisseurs étrangers qui cherchent à en prendre le contrôle. Je pense notamment à l’entreprise Latecoere dernièrement. Afin de répondre aux inquiétudes des entreprises du secteur et particulièrement des PME et TPE, le Sénat avait voté la création d’un livret souveraineté lors de l’examen de la loi de programmation militaire, l’été dernier. paritaire (CMP), un accord avait été trouvé pour que soit fléchée vers ces entreprises une partie des ressources du livret A et du livret de développement durable et solidaire. à la faveur de l’examen d’un recours de députés d’opposition concernant la loi de programmation militaire, le Conseil constitutionnel s’est saisi d’office d’une dizaine d’articles. Ces derniers ont été censurés au titre de l’article 45 de la Constitution. Ce fut notamment le cas de l’article 52 portant sur le financement de ces entreprises de la défense.

C’est pourquoi, madame la ministre, cette proposition de loi nous paraît pertinente et nécessaire pour soutenir cette filière d’excellence au service de l’indépendance de notre BITD et de notre souveraineté nationale.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà plus de deux ans que l’Europe connaît de nouveau la guerre sur son sol. Plus de deux ans pendant lesquels la France est venue en aide à l’Ukraine en lui fournissant un appui matériel, dont l’impact économique pour notre pays n’est pas négligeable. Nous réalisons aujourd’hui le retard immense accumulé par la France dans le financement de ses armées et de leurs équipements, et ce dans un contexte d’économie de guerre. Les auteurs de la proposition de loi que nous examinons ont cherché à dégager des solutions concrètes pour rattraper, au moins en partie, notre retard. texte est la meilleure des solutions d’attente, celle qui peut nous permettre d’effectuer la meilleure transition possible vers un modèle plus durable d’économie de la défense. Fruit du travail de notre collègue Pascal Allizard et de l’expertise conjointe des deux commissions concernées, loi vise à apporter, immédiatement, une première réponse à nos difficultés structurelles de financement. Plus que jamais, nos entreprises de défense, majoritairement des PME, doivent changer de modèle économique. Elles doivent monter en cadence pour faire face à la demande croissante, seulement au conflit ukrainien, mais également aux besoins futurs de notre pays, dans l’éventualité où cette guerre viendrait malheureusement à se généraliser. L’esprit de ce texte est largement détaillé dans son article 1 : il s’agit de dépasser les problématiques de nos entreprises que constituent le manque de fonds propres et la dépendance aux exportations. Dans un contexte de réarmement de l’Union européenne face aux nouvelles menaces, les auteurs de la proposition de loi entendent garantir le financement, et donc la souveraineté, de nos pépites technologiques de défense. L’article 1 prévoit ainsi la possibilité de fléchage d’une partie des ressources collectées au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire vers le financement des PME et entreprises de taille intermédiaire de la BITD. Portée de manière Portée de manière transpartisane, et adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation militaire, cette mesure indispensable avait pourtant été censurée par le Conseil constitutionnel,

afin non seulement d’appréhender son efficacité, mais également de réfléchir à l’opportunité de mettre en place un produit d’épargne spécifique dédié au financement des entreprises de défense. Sur proposition du rapporteur de la commission des finances, la date de remise de ce rapport a été avancée d’un an afin de maintenir l’écosystème sous tension. Il est en effet absolument indispensable d’avancer rapidement dans ce domaine : plus nous attendrons, plus nous serons exposés aux conséquences d’un financement inadapté. Mes chers collègues, ce texte est gage de sagesse. Il l’est d’autant plus au moment où certains cherchent, à dessein ou non, à nous engager toujours plus avant dans une démarche cobelligérante qui nous serait fatale. Au moment où le conflit ukrainien entre dans une nouvelle phase, cette proposition de loi constitue un apport direct et efficace à la loi de programmation militaire, que nous avons largement adoptée l’année dernière. Elle permettra, en complémentarité avec cette dernière, d’inciter au mieux nos entreprises, les acteurs publics et les partenaires privés à avancer main dans la main pour assurer la pérennité de la défense française. Telle est la condition pour préserver notre souveraineté face aux nouvelles menaces extérieures qui affectent notre pays ! La discussion

et qu’il fallait trouver d’autres façons de financer l’effort de défense. Une fois n’est pas coutume, je partage l’avis du ministre. Le texte prévoit désormais de modifier le fléchage des encours non centralisés du livret A et du livret de développement durable et solidaire. Malgré cela, j’estime que la philosophie première du livret A doit être maintenue : celui doit continuer à financer exclusivement les besoins sociaux et écologiques, conformément à sa vocation première, dans un contexte où la lutte contre le dérèglement climatique n’est pas à la hauteur des enjeux et où la crise du logement s’aggrave. Aujourd’hui, ce sont plus de 4 millions de Français qui souffrent quotidiennement du mal logement. Sur la dernière décennie, le nombre de ménages demandeurs de logements sociaux a augmenté de plus d’un million, alors que l’offre de HLM disponibles est restée relativement stable. Par ailleurs, ces chiffres, qui reflètent la crise alarmante du logement, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui vivent dans la promiscuité. Ma position est claire, mes chers collègues : pas le moindre centime ne doit manquer pour venir en aide à nos concitoyens qui peinent à se loger dignement. J’irai même plus loin : l’effort n’est pas suffisant Par ailleurs, concernant le dérèglement climatique, les fonds et les efforts sont, là aussi, loin d’être suffisants. Pourtant, nous savons pertinemment que la transition écologique nécessite de mobiliser le maximum de moyens pour financer les actions nécessaires. Je ne nie ni les difficultés et le besoin de financement que rencontrent certaines petites et moyennes entreprises du secteur de la défense ni le caractère hautement stratégique de celles ci pour la Nation. Mais d’autres pistes existent. Penchons nous, par exemple, mes chers collègues, sur la chaîne de valeur dans l’industrie de défense ou réfléchissons

uns : 4,2 millions de personnes non ou mal logées ; 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement ; 1 million de personnes vivant en habitat indigne ; 2,5 millions de ménages en attente d’un logement social. Voilà ce dont nous devrions parler à la faveur d’une proposition de loi qui concerne le livret A. Voilà l’urgence qui frappe notre pays.

nous nous apprêtons aujourd’hui à ponctionner l’épargne des Français pour une industrie qui bénéficie par ailleurs de largesses inégalées de la part de l’État et de ses opérateurs, comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale. C’est pour éviter cette flibusterie visant l’épargne populaire que nous vous proposons de supprimer l’article 1 de cette

Premièrement, un livret spécifique ne collecterait sans doute pas suffisamment d’argent. De ce fait,

le soutien à l’Ukraine, ce que l’on peut entendre. En effet, si l’Ukraine tombe, c’est l’Europe entière qui sera menacée par le boucher de Russie. Les milliers de soldats ukrainiens et de volontaires internationaux qui se battent sans relâche nous défendent aussi, et pour qu’ils gagnent, il faut les soutenir, avec du matériel, de l’équipement, de l’armement.

pour une durée de deux ans. Ce rendez vous permettra au législateur de considérer la situation sur le front ukrainien pour décider s’il y a lieu, ou non, de poursuivre ce dispositif.

blanc de la défense, l’identification des acteurs de la base industrielle et technologique de défense reste difficile. En tout état de cause, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne permet pas de faire la lumière sur les entreprises susceptibles de bénéficier des financements issus de l’épargne populaire.

En effet, il ne suffit pas de se revendiquer comme un acteur de la BITD pour être réellement une entreprise industrielle de défense. C’est l’un des nombreux griefs que nous formulons envers cette proposition de loi et que nous vous proposons de corriger.

S’il paraît évident que Bercy détermine cette part, notamment parce que tout ce qui n’est pas affecté au financement de la BITD bénéficie au reste de l’économie, il nous semble en revanche opportun que le ministère des armées puisse également faire remonter les besoins spécifiques de ce secteur d’activité, notamment au regard de la loi de la loi de programmation militaire. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui vise à prévoir que la détermination de la fraction affectée aux entreprises de la BITD sera déterminée non par un arrêté du seul ministre chargé de l’économie, mais par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des armées.

Ainsi que je l’ai rappelé précédemment, si le fléchage de ces encours vers le financement des entreprises de la défense ne résoudra pas l’ensemble de leurs difficultés de financement, il constitue néanmoins un signal politique clair en faveur de ces entreprises. Nous devons signifier aux acteurs financiers

n’ont pas été de nature à me convaincre. Permettez moi de citer un passage du rapport : « Ainsi que l’ont rappelé l’ensemble des acteurs entendus par le rapporteur, les entreprises de l’industrie de défense française se heurtent tout d’abord aux mêmes difficultés de financement bancaire que celles rencontrées par l’ensemble des entreprises françaises. Leurs marges sont faibles, et leurs investissements aussi, tout comme leur pouvoir de marché. Pour autant, les banques françaises figurent parmi les plus actives au niveau mondial dans le domaine de la défense.

Plus loin, le rapport nous apprend que « les quelques cas de refus de crédit bancaire opposé à des entreprises de l’industrie de défense française ne trouvaient pas principalement leur origine dans leur secteur d’activité, mais dans leur situation financière. Par ailleurs, si le secteur de la défense n’apparaît pas en tant que tel dans les statistiques sectorielles de la Banque de France et de la médiation du crédit, il convient de relever qu’aucun d’entre eux n’a relevé de biais en défaveur des industries de ce secteur. » Les arguments invoqués pour justifier de difficultés de financement des PME du secteur de la défense ne sont donc pas viables.

Si cette médiation n’aboutissait pas, ce qui est le cas seulement quatre fois sur dix, alors l’épargne des Français pourrait financer, en dernier recours, si je puis dire, les entreprises industrielles de défense.

Pour lutter contre les menaces informationnelles, pour se protéger contre les cyberattaques, pour bâtir des stratégies d’influence, pour sécuriser l’approvisionnement énergétique, des entreprises issues d’autres secteurs d’activité peuvent aussi contribuer utilement au renforcement de la souveraineté nationale.

les banques font en effet preuve d’une grande frilosité lorsqu’il s’agit de leur accorder des prêts. C’est d’ailleurs l’une des raisons de notre présence dans cet hémicycle aujourd’hui.

L’industrie française de défense et, plus largement, l’industrie européenne de défense soutiennent que les entreprises de la BITD devraient être explicitement incluses dans la catégorie des activités durables, afin de préserver les voies de financement auxquelles elles auraient accès. Soutenues par les ministres de la défense de l’Union dans une déclaration commune le 14 novembre dernier, ces industries demandent depuis longtemps davantage d’indulgence quant à la mise en œuvre des critères ESG. Nous estimons, pour notre part, que la base industrielle et technologique de défense européenne joue un rôle indispensable dans la sûreté et la sécurité globale de l’Europe. Financer nos entreprises européennes, c’est rendre véritablement crédible notre capacité à contribuer à la paix, à la stabilité et à la durabilité sur notre continent. Par cet amendement, nous demandons donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’accès des entreprises françaises de la BITD au financement européen.

de la proposition de loi. En effet, l’ensemble des établissements bancaires doivent déjà rendre compte de la façon dont ils satisfont aux objectifs fixés par le législateur quant au fléchage des encours non centralisés du livret A.

à convaincre mon ministre de tutelle et le ministre des armées qu’il fallait nous engager pour passer d’un avis de sagesse à un avis favorable sur cet amendement

Dont acte. Madame la ministre, si tel était le cas, pourquoi ne pas avoir obligé les banques à financer nos entreprises de la base industrielle et technologique de défense,

vous avez soulevé. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 13 mars, l’après midi, d’une déclaration, suivie d’un débat et d’un vote, en application de l’article 50 50 1 de la Constitution, relative au débat sur l’accord de sécurité franco ukrainien et la situation en Ukraine. Acte est donné de cette demande. Cette déclaration interviendrait après le débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. Nous pourrions prévoir que les orateurs des groupes, à raison d’un orateur par groupe, interviennent, selon l’ordre décroissant de leur effectif, avec les temps de parole suivants : quatorze minutes pour le groupe Les Républicains ; douze minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dix minutes pour le groupe Union Centriste ; huit minutes pour les autres groupes ; trois minutes pour un sénateur non inscrit. Le délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat serait fixé au mardi 12 mars, à quinze heures. Y a t il des observations ?… Il en est ainsi décidé. En conséquence, le temps de parole des orateurs pour le débat sur le rapport de la Cour des comptes serait fixé à quarante nous pourrions prévoir la suite de l’examen de la proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative le jeudi 14 mars, en premier point de l’ordre du jour. Y a t il des observations ?…